En application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, ainsi que de la loi organique n° 2010-837 et de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 prises pour son application, la commission de l'aménagement du territoire a émis, lors de sa réunion de ce jour, un avis favorable- 19 voix pour, 9 voix contre -à la reconduction de M. Augustin de Romanet aux fonctions de président-directeur général de la société Aéroports de Paris. Par ailleurs, conformément aux mêmes dispositions, la commission des affaires étrangères a émis un avis favorable à la reconduction de M. Rémy Rioux- 24 voix pour, 3 voix contre, 8 bulletins blancs -aux fonctions de directeur général de l'Agence française de développement. L'ordre du jour appelle la nomination des 21 membres de la mission d'information sur la sous-utilisation chronique des fonds européens en France, créée à l'initiative du groupe les Indépendants-République et Territoires, en application du droit de tirage prévu par l'article 6 du règlement.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 L'ordre du jour appelle l'examen de deux projets de loi tendant à autoriser la ratification ou l'approbation de conventions internationales. Pour ces deux projets de loi, la conférence des présidents a retenu la procédure d'examen simplifié. Je vais donc les mettre successivement aux voix. Je mets aux voix le texte adopté par la commission sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord-cadre relatif à la coopération en matière de sécurité sanitaire entre le Gouvernement de la République française et la Principauté de Monaco

armées est favorable à l'adoption de ce texte. Je mets aux voix le texte adopté par la commission sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Arménie

armées est favorable à l'adoption de ce texte. L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions des commissions mixtes paritaires chargées d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique

un accord sans aucune difficulté. Cette heureuse conclusion est l'aboutissement d'untravail mené en étroite concertation avec toutes les le Gouvernement, bien sûr, mais aussi chacune desdeux assemblées, ainsi que les parlementaires polynésiens, que je salue, lesreprésentants des institutions de la Polynésie française et tous ceux qui se sentent concernés par l'avenir de ce beau territoire. Je veux remercier très sincèrement Mme la ministre des outre-mer et mon homologue rapporteur de l'Assemblée nationale, Guillaume Vuilletet, de ce travail constructif. Ces deux textes visent pour l'essentiel à moderniser le statut de la Polynésie française pour faciliter l'exercice de ses compétences par le pays, ainsi que sa coopération avec l'État et les communes polynésiennes. Alors que les précédentes révisions du statut, en 2007 et en 2011, avaient plutôt pour objet de resserrer la réglementation pour mettre fin aux dérives observées par le passé, la réforme actuelle est un témoignage de confiance à à l'égard des responsables polynésiens, qui ont su renouer avec la stabilité institutionnelle, assainir la situation budgétaire du pays et remettre son économie en marche. Le projet de loi organique a également pour objet decorriger une malfaçon de la réforme de 2011 en ce quiconcerne les modalités de remplacement des représentants à l'assemblée de la Polynésie française. Il est urgent demettre fin à une incertitude juridique qui met en péril lastabilité des institutions du pays. Enfin, le projet de loi organique reconnaît solennellement la contribution, ou plutôt la mise à contribution, de la Polynésie française pour la construction de la capacité de dissuasion nucléaire et la défense de laNation. Il inscrit en tête du statut de la Polynésie les principesde l'indemnisation des victimes des essais nucléaires, del'entretien et de la surveillance par l'État des sitesd'expérimentation et de l'accompagnement de la reconversionéconomique et structurelle du pays à la suite de la fin des essais. Ces dispositions, je le sais, répondent à une attente fortede nos concitoyens polynésiens et traduisent dans la loiorganique les engagements pris par l'État dans le cadre del'accord de Papeete du 21 février 2017. En première lecture, le Sénat a enrichi très substantiellement les deux textes, pour répondre mieux aux besoins de la Polynésie. J'en veux pour preuve la réforme du régime contentieux des lois du pays, qui permettra d'accélérer la mise en oeuvre des politiques locales, la nouvelle faculté donnée aux autorités polynésiennes de saisir le Conseil d'État de questions de droit portant sur la délimitation de leurs compétences et sur le domaine des lois du pays, l'assouplissement du régime des sociétés publiques locales, les SPL, créées par la Polynésie française, ainsi que des incompatibilités frappant les membres d'autorités administratives indépendantes locales, la transformation de la dotation globale d'autonomie en prélèvement sur recettes, afin de sanctuariser cette ressource versée à la Polynésie française depuis la fin des essais nucléaires et destinée à accompagner sa reconversion, l'ajout de dispositions visant à encourager la coopération entre les collectivités polynésiennes ou encore d'importantes dispositions, inspirées de la proposition de loi du député Serge Letchimy, visant à faciliter la sortie de l'indivision foncière en Polynésie

qui ont contribué à la rédaction de la partie du rapport consacrée au foncier. Nos collègues députés, constatant que les deux textes étaient parvenus à un équilibre, n'y ont apporté que des modifications légères, mais utiles. Outre diverses retouches rédactionnelles, l'Assemblée nationale a ainsi précisé la portée de plusieurs dispositions et les a complétées en supprimant l'extension, malvenue en Polynésie française, de la dépénalisation du stationnement payant. En commission mixte paritaire, il ne nous restait donc qu'à opérer quelques corrections de pure forme, ainsi qu'une coordination avec la loi tendant à sécuriser l'actionnariat des entreprises publiques locales, due à l'initiative de notre collègue collègue Hervé Marseille, qui vient d'être adoptée dans les mêmes termes par les deux assemblées. Nous avons par ailleurs confirmé la suppression de deux demandes de rapport, portant respectivement sur l'accessibilité et l'intelligibilité du droit en Polynésie française et sur le placement de leurs fonds libres par le pays et ses établissements publics. Je sais que notre collègue Lana Tetuanui en a conçu quelques regrets, mais je veux la rassurer : plutôt que de demander au Gouvernement des rapports qui ne viendront jamais, le Parlement se saisira lui-même de ces questions, notamment de celle de celle de l'intelligibilité du droit applicable en Polynésie française et dans les autres collectivités ultramarines. J'ai pu mesurer, en travaillant sur le projet de loi ordinaire, combien il est difficile pour toute personne normalement constituée de comprendre certaines dispositions d'adaptation du droit en Polynésie. Ce n'est pas un hasard si les Polynésiens appellent le code général des collectivités territoriales, le CGCT, le code général « casse-tête » ! Il faut y réfléchir réfléchir sérieusement, d'autant que le problème pourrait bientôt se généraliser avec les progrès de la différenciation territoriale. Je sais aussi que certains auraient souhaité que nous allions encore plus loin dans la rénovation du statut de la Polynésie française et dans la compensation des dommages provoqués par les essais nucléaires sur ce territoire. Nous avons fait ce qu'il était possible de faire, dans le cadre de la loi organique ou ordinaire et dans le respect de la Constitution. Nous resterons vigilants globale d'autonomie, la DGA, en prélèvement sur recettes et sur la manière dont elle sera traduite dans la prochaine loi de finances. En tout état de cause, je veux que chacun mesure les avancées que comprennent ces deux projets de loi, à l'issue de la navette parlementaire. Demain, grâce à ces deux textes, les institutions de la Polynésie française seront plus solides, leur fonctionnement sera plus fluide, les problèmes fonciers rencontrés

Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, je ne vous cache pas que je suis, à la fois, heureuse de finaliser le travail de grande qualité que nous avons mené conjointement sur ces projets de loi organique et ordinaire relatifs au statut d'autonomie de la

le travail de ces deux années montre que la majorité, le Président de la République, Emmanuel Macron, et le Gouvernement se sont inscrits dans la continuité de l'État sur ce dossier. En effet, je le rappelle, ces textes sont le pendant législatif de l'accord de l'Élysée, signé le 17 mars 2017, 2017, qui a marqué le renouveau des relations entre l'État et la Polynésie française. En reconnaissant le fait nucléaire et ses conséquences, la Nation a adressé un message symbolique très fort à la Polynésie française, qui n'élude pas la réalité des faits. L'indemnisation des victimes des essais nucléaires va bien entendu se poursuivre, et la mémoire des Polynésiennes et des Polynésiens sera sanctuarisée, notamment par le centre de mémoire, pour lequel l'État a transféré du foncier à titre gratuit. Je renouvelle mes titre gratuit. Je renouvelle mes chaleureux remerciements à la sénatrice Lana Tetuanui, qui, vous le savez, a largement oeuvré pour que ces dispositifs aboutissent. Je n'oublie pas, bien sûr, son collègue Nuihau Laurey, qui a participé aux nombreux échanges entre le ministère des outre-mer et

Comme vous pouvez le constater, le Gouvernement a tenu ses engagements, puisque la rédaction proposée par la sénatrice Lana Tetuanui n'a pas bougé d'un iota.

est la condition pour faire rayonner les outre-mer à la hauteur des ambitions que nous leur assignons. Permettez-moi de remercier singulièrement l'ensemble des groupes politiques de votre assemblée

ministre ont tout dit. Ces deux textes, attendus depuis plusieurs années, sont le fruit d'échanges anciens, nourris et riches entre les élus de Polynésie française, la ministre des outre-mer et les commissions des lois du Sénat et de l'Assemblée nationale. C'est d'ailleurs cet esprit de concorde qui a prévalu durant nos travaux et lors de la navette parlementaire, puisque les modifications apportées par l'Assemblée nationale ont largement conservé les équilibres auxquels nous étions parvenus.

C'est donc, encore et toujours, cet esprit de coopération, dans la lignée de celui des accords de l'Élysée du 17 mars 2017, signés par François Hollande et Édouard Fritch, qui a concouru, le 7 mai dernier, à l'aboutissement de la commission mixte paritaire. Cela a été rappelé, les deux textes dont l'examen nous réunit aujourd'hui procèdent au toilettage statutaire et institutionnel du statut de la Polynésie française qui s'imposait pour faciliter l'exercice des compétences du pays et sa coopération avec l'État et les communes. En outre, le projet de loi organique reconnaît solennellement la dette nucléaire de la France envers la Polynésie française. Quant au projet de loi ordinaire, il contient des dispositions, auxquelles j'attache une importance toute particulière, sur la sortie de l'indivision, laquelle stérilise une grande partie du foncier disponible, non seulement en Polynésie, mais également partout ailleurs en outre-mer. Issues du rapport d'information du 23 juin 2016, fait au nom de la délégation sénatoriale aux outre-mer, sur la sécurisation des droits fonciers dans les outre-mer, elles faciliteront grandement, j'en suis persuadé, la vie des Polynésiens. Je salue également la sanctuarisation de la dotation globale d'autonomie de la Polynésie française, transformée en prélèvement sur recettes en 2020. Je tiens à féliciter, à mon tour, nos collègues polynésiens Lana Tetuanui et Nuihau Laurey,

Mes chers collègues, vous l'aurez compris, le groupe La République En Marche votera en faveur de l'adoption de ces deux textes, qui marquent la volonté du Gouvernement d'entretenir une relation de confiance avec les autorités polynésiennes et sont porteurs d'avancées réelles pour nos compatriotes polynésiens.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, débutés il y a quelques mois, nos travaux visant à réformer le statut d'autonomie de la Polynésie française touchent à leur fin. Une fois n'est pas coutume, l'Assemblée nationale et sa majorité présidentielle ont accepté de jouer le jeu du compromis parlementaire en soutenant nombre d'apports constructifs issus du Sénat et en permettant à la commission mixte paritaire d'aboutir positivement. C'est à saluer. La Polynésie française méritait bien un tel sens des responsabilités. Nous avons toutes et tous eu l'occasion de le rappeler en première lecture, la situation dans ces territoires ultramarins est préoccupante. Avec ses 24 % de chômeurs, son climat propice aux catastrophes naturelles et ses services publics défaillants, cette collectivité d'outre-mer a besoin d'une transformation profonde de ses statuts. Cette réforme promise aux Polynésiens, qui ont été consultés préalablement à la rédaction du projet de loi et du projet Évidemment, nous soutenons le nouvel acte de décentralisation qui entraîne un réajustement équilibré des compétences entre l'État et les institutions polynésiennes, puisque Paris ne peut exercer convenablement son administration au sein des territoires polynésiens à à près de 20 000 kilomètres de distance. De même, nous saluons les mesures visant à redynamiser le dialogue social et le tissu économique local. En somme, ces textes de loi ont pour objet de rendre le droit appliqué en Polynésie plus lisible et de permettre une gouvernance de ces territoires plus proche et plus adaptée aux besoins des habitants de l'archipel. Mais, en tant qu'élue écologiste, je ne peux que regretter le manque de courage du Gouvernement et de la droite sénatoriale De nombreux amendements substantiels allant dans le sens de la protection de l'environnement vous ont été soumis en première lecture, tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, par les divers groupes de gauche. Tous ont été rejetés. Je ne peux m'empêcher de m'interroger : pourquoi une telle frilosité ? À l'heure de la sixième extinction de masse des espèces vulnérables, la préservation du patrimoine naturel polynésien est un enjeu majeur. La Polynésie française ne peut être appréhendée si l'on ne reconnaît pas la dimension hautement culturelle et sociale qui lie ses habitants à son environnement et à ses ressources naturelles. De ce fait, nous aurions pu espérer un soutien renforcé de l'État dans la protection de la biodiversité des récifs coralliens polynésiens, notamment dans le cadre de l'exploitation commerciale des terres rares. Des dispositions venant renforcer la lutte contre la pêche illégale et la surpêche industrielle vidant nos océans auraient également été nécessaires. La zone économique exclusive polynésienne s'étend en effet sur 5,5 millions de kilomètres carrés. Les eaux polynésiennes sont riches en poissons et attirent de nombreuses flottilles étrangères qui violent nos eaux territoriales. Face à ces activités, préserver la biodiversité marine, si chère à la Polynésie, est une responsabilité de l'État français. Nous déplorons également qu'aucune mesure n'ait été adoptée en faveur d'une protection accrue des plages locales. À l'échelle mondiale, sur les 275 millions de tonnes de plastiques produits, près de 10 millions finissent dans les océans. À ce rythme, à l'horizon 2050, il y aura davantage de déchets plastiques que de poissons dans les fonds marins Ce phénomène pourrait avoir des répercussions dramatiques sur la santé humaine et animale. Pour preuve, 100 000 animaux, notamment des tortues et des oiseaux de mer, sont tués par les plastiques chaque année. Une plus grande vigilance dans ce domaine relève de l'urgence. Enfin, au regard du climat nettement tropical des outre-mer, nous avions les moyens de devenir les champions des énergies propres, notamment hydraulique et solaire, et ainsi de pallier la fin du nucléaire énergétique polynésien. Une telle transition ne semble pourtant pas être une priorité pour l'exécutif. Mes chers collègues, il faut reconnaître que ces deux textes présentent des lacunes. Mais ils constituent également, dans leur ensemble, une avancée législative relativement importante importante et prometteuse. Les Polynésiens ont besoin d'un droit plus clair, plus adapté, d'une économie plus sociale et florissante, d'un environnement plus sain et préservé.

de la réussite des deux commissions mixtes paritaires, réunies en une seule, qui ont approuvé le bon compromis dû au travail des rapporteurs, et tout particulièrement de celui du Sénat, M. Darnaud.

La République reconnaît la mise à contribution de la Polynésie française pour la construction de la capacité de dissuasion nucléaire et la défense de la Nation. » Cette formulation est tout à fait judicieuse

aura pour effet de la pérenniser, ce qui est important pour le financement de la Polynésie française. D'autres mesures techniques ont été approuvées lors de la commission mixte paritaire,

De même, Thani Mohamed Soilihi l'a dit, les mesures pour lutter contre l'indivision foncière sont précieuses,

Comme je l'avais alors souligné lors de la discussion générale, ces deux textes s'inscrivent dans une phase de normalisation des rapports avec la métropole pour les collectivités concernées par l'article 74 de notre Constitution. 74 de notre Constitution. Il n'est pas inutile de rappeler à ce stade que mon territoire, Saint-Martin, dix ans après son accession au statut de collectivité d'outre-mer, se doit d'accentuer sa réflexion vue d'une indispensable modernisation et adaptation de son statut actuel aux nouvelles exigences que lui impose une société en perpétuel mouvement et mutation. Lors de l'examen de ces textes en février, notre groupe, le RDSE, n'avait émis que quelques réserves. Nous nous étions tout d'abord interrogés sur les dispositions relatives aux autorités administratives indépendantes, comme nous le faisons systématiquement, s'agissant de ces organismes, depuis le rapport de notre excellent ancien collègue Jacques Mézard. Suivant la même logique, il nous avait semblé cohérent de rappeler les dispositions contenues dans la loi pour le pour le développement des sociétés publiques locales, adoptée en 2010, qui fixaient comme exigence le maintien d'une présence obligatoire de deux actionnaires au minimum, alors que l'article 5 du texte ouvre la possibilité d'un actionnaire unique.

de nous prononcer, il convient donc d'examiner les points de divergence qui ont été traités. Pour le projet de loi organique, seul l'article 1 posait question. Bien que de faible portée normative, cet article est très attendu par les Polynésiens, car il traite de la question sensible des essais nucléaires. Après les déclarations faites par le président François Hollande en 2016, reconnaissant les conséquences sanitaires et environnementales de ces essais, et un long processus de mûrissement et de concessions réciproques, cet article 1 vient aujourd'hui concrétiser cette reconnaissance. Il est donc indispensable qu'il soit maintenu dans le texte. Afin de surmonter la petite divergence entre les deux assemblées,

Les articles 14 et 16, qui étaient des demandes de rapport, ont été supprimés. En somme, la commission mixte paritaire a essentiellement entériné des modifications de la rédaction de plusieurs articles sans changer substantiellement les deux textes. textes. En ce moment tant attendu par la population et les élus polynésiens, et avant le vote définitif de notre assemblée, il ne me semble pas superflu d'adresser une fois de plus nos remerciements à Mme la ministre,

Le RDSE, de façon unanime et conformément à son vote de février dernier, apporte son soutien aux Polynésiens, qui expriment clairement leur volonté de poursuivre leur marche en avant, tout en montrant leur attachement à la République. Mes collègues et moi-même exprimons notre fierté d'avoir participé à ces débats de qualité, qui se sont conclus par un vote quasiment unanime en première lecture ; nous devrions parvenir aujourd'hui au même résultat. La parole

en l'absence de nos collègues polynésiens, j'ai l'honneur et le plaisir d'intervenir aujourd'hui sur les deux projets de loi se rapportant à la Polynésie française, collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution. Ces projets de loi, déposés sur le bureau du Sénat le 12 décembre 2018, examinés en première lecture le 13 février 2019 et adoptés à l'unanimité par notre assemblée, puis modifiés et votés à l'Assemblée nationale le 11 avril, ont fait l'objet d'une commission mixte paritaire conclusive le 7 mai dernier. Nous nous en félicitons. Cette loi organique et cette loi simple, qu'il nous appartient aujourd'hui d'entériner, visent à moderniser le statut de la Polynésie française pour faciliter l'exercice de ses compétences par le pays ainsi que sa coopération avec l'État et les communes. Je suis heureux que ces textes satisfassent dans une large la volonté de la majorité gouvernementale du pays de la Polynésie française et concrétisent un engagement fort de la République à l'égard de cette collectivité d'outre-mer marquée par le fait nucléaire. En effet, outre l'impératif de modernisation de la loi statutaire, cette réforme élève au rang législatif la reconnaissance du fait nucléaire et de toutes ses incidences économiques, sanitaires et environnementales, qui ont profondément marqué la société polynésienne.

à un voeu très cher des Polynésiens et constitue un acte ayant valeur de « pacte de confiance », qu'il convenait de sanctuariser dans la loi statutaire. Le voeu des élus polynésiens était également d'aller plus loin dans la sanctuarisation de la dotation globale d'autonomie, dite « dette nucléaire

qui déterminera de manière pérenne le montant de la dotation globale d'autonomie, conformément aux engagements de l'État pris en 1996 lors de l'arrêt des essais nucléaires. Il conviendra donc de veiller à opérer ce prélèvement sur recettes au travers de la prochaine loi de finances. Par ailleurs, il était essentiel de toiletter le statut de large autonomie dont bénéficie la Polynésie, pour un fonctionnement plus efficient de ses institutions et dans une perspective de développement économique durable. À ce titre, permettez-moi de faire un peu d'histoire, pour rappeler les grandes dates ayant jalonné le parcours menant au statut d'autonomie de la Polynésie française. Cette marche de la Polynésie vers l'autonomie est ancienne. Établissement français de l'Océanie à l'origine, devenu territoire d'outre-mer dénommé « Polynésie française » en 1957, ce territoire a connu de nombreuses réformes statutaires visant à répondre aux attentes légitimes des élus locaux en matière de gestion de leurs propres affaires. Ainsi, dès 1977, une première tentative d'autonomie de gestion avait été mise en oeuvre, mais ce n'est qu'en 1984 qu'une véritable autonomie dite « interne » a été concédée au territoire de la Polynésie. En 1996, c'est la loi organique du 1 avril qui conféra à la Polynésie un nouveau statut d'autonomie, avec une personnalité propre et des compétences accrues, au moment même où s'interrompaient les essais nucléaires. Enfin, en 2004, c'est par l'adoption de la loi organique du 27 février que la Polynésie française devient un pays d'outre-mer. Elle dispose donc désormais d'une très large autonomie : il est clairement prévu que « la Polynésie se gouverne librement et démocratiquement par ses représentants élus et par la voie du référendum local ». Après plus d'une décennie d'application de la loi organique de 2004, il convenait d'améliorer, de toiletter ce statut, et de clarifier certaines de ses dispositions. C'est l'objet des deux textes présentés par le Gouvernement, que de nombreux amendements du Sénat puis de l'Assemblée nationale sont venus enrichir. On relèvera néanmoins, pour la regretter, la suppression de deux rapports, prévus aux articles 14 et 16 du qui avaient pourtant fait l'objet d'un accord et d'un engagement de Mme la ministre lors de la première lecture au Sénat. L'essentiel des réformes prévues par ces deux projets de loi vont toutefois, heureusement, permettre notamment d'introduire une plus grande stabilité politique grâce à la correction de l'anomalie de l'article 107 relatif aux modalités de remplacement des représentants à l'assemblée de Polynésie

du régime contentieux des lois de pays afin d'accélérer la mise en oeuvre des politiques publiques locales, des adaptations du code civil spécifiques à la Polynésie, très importantes pour tenter de régler au mieux l'indivision successorale, de nombreuses adaptations du code général des collectivités territoriales pour ce qui concerne les communes et la parité au Conseil économique, social, et culturel et environnemental.

Je tiens également à remercier, au nom de mon groupe et particulièrement de ses membres polynésiens, notre collègue Mathieu Darnaud et le député Guillaume Vuilletet, qui ont su appréhender les attentes de la Polynésie française et mesurer pleinement les spécificités de ce territoire. Enfin, je remercie Mme la ministre de son écoute et sa disponibilité tout au long de nos travaux. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, le groupe Union Centriste votera bien entendu ces deux projets de loi en faveur de la modification du statut de la Polynésie française,

stratégiques, géographiques et culturels, ainsi qu'en termes de biodiversité. C'est une longue histoire qui lie la France et la Polynésie- pays d'outre-mer « au sein de la République » -dans un destin commun, et les deux textes qui nous ont été soumis s'inscrivent dans ce contexte. L'actuel statut de la Polynésie française avait été révisé en 2007 et en 2011. Depuis plusieurs années, des ajustements étaient attendus. Ils ont fait l'objet de négociations approfondies qui ont abouti à la signature des accords de l'Élysée, le 17 mars 2017. Ces deux textes en sont la traduction législative. Ils visent, pour l'essentiel, à moderniser le statut de la Polynésie française pour faciliter l'exercice de ses compétences par le pays, ainsi que sa coopération avec l'État et les communes polynésiennes. Le projet de loi organique a notamment pour objet de corriger un défaut de la réforme de 2011, relatif aux modalités de remplacement des représentants à l'assemblée de la Polynésie française. Cette disposition, qu'il était urgent de prendre, permet de remédier au risque d'instabilité institutionnelle du pays. Il reconnaît également, de façon solennelle, l'immense contribution de la Polynésie française à la construction de la capacité de dissuasion nucléaire et à la défense de la Nation. Il inscrit en tête du statut de la Polynésie les principes de l'indemnisation des victimes des essais nucléaires, de l'entretien et de la surveillance par l'État des sites d'expérimentation et de l'accompagnement de de la reconversion économique et structurelle du pays à la suite de la fin des essais. Je me réjouis que le travail parlementaire ait permis d'enrichir très substantiellement les deux textes. Je citerai en particulier la réforme du régime contentieux des lois du pays, qui permettra d'accélérer la mise en oeuvre des politiques locales, la faculté donnée aux autorités polynésiennes de saisir le Conseil d'État de questions de droit portant sur la délimitation de leurs compétences et sur le domaine des lois du pays, ou encore l'assouplissement du régime des sociétés publiques locales créées par la Polynésie française,

versée à la Polynésie française depuis la fin des essais nucléaires et destinée à accompagner sa reconversion. Je veux enfin mentionner les dispositions visant à encourager la coopération entre les collectivités polynésiennes, ou encore les mesures qui faciliteront la sortie de l'indivision foncière. Avant de conclure, je souhaite remercier Mme la ministre

Madame la ministre, mes chers collègues, l'Océanie et la France partagent une histoire multiséculaire. Ces deux projets de loi, organique et ordinaire, sont fondamentaux pour la Polynésie car ils lui donnent davantage de moyens institutionnels pour construire son avenir avec confiance et reconnaissent solennellement la « dette nucléaire » de la République à son égard. Le groupe Les Indépendants votera en faveur de l'adoption de ces deux textes qui réaffirment la place de la Polynésie dans l'histoire et le fonctionnement de notre République.

Monsieur le président, madame la ministre, chers collègues, je me félicite du changement d'état d'esprit qui a présidé à ces textes marqués, comme l'a fort pertinemment relevé notre collègue rapporteur, Mathieu Darnaud, par la confiance. Cela permet de tourner le dos à une période d'encadrement et de régulation institutionnelle. C'est le signe du bon fonctionnement des institutions de la Polynésie française, qui peuvent ainsi se tourner vers l'avenir avec sérénité ; je m'en réjouis, naturellement. Il n'est un secret pour personne ici que je suis un fervent partisan de la différenciation territoriale, dont la confiance est un des fondements. Je suis en effet profondément convaincu que l'efficience passe par une meilleure adéquation aux réalités par une contextualisation des mesures, en laissant les collectivités agir chaque fois que cela est possible, car elles sont au plus près de leurs réalités. Dans cette optique, l'État doit accompagner les collectivités locales et leur garantir une véritable autonomie afin qu'elles puissent la mettre au service de leur développement endogène. Les textes que nous examinons aujourd'hui ont été élaborés conjointement avec les élus locaux, ce qui nous apporte la meilleure preuve qu'ils correspondent à la volonté locale. C'est encore un point de satisfaction. aurait pu sans difficulté faire référence au « renforcement du statut de la Polynésie française ». Pour en terminer avec ces quelques considérations d'ordre général, je tiens à souligner l'expertise de notre collègue Mathieu Darnaud et à saluer la qualité de son travail.

Je me contenterai d'évoquer les quelques dispositions qui ont plus particulièrement retenu mon attention. En premier lieu, il est important que la loi soit la traduction fidèle de la reconnaissance de la place de la Polynésie française dans la construction de la capacité de dissuasion nucléaire de la France. Ainsi, se borner à affirmer sa contribution au processus de construction de force nucléaire sans reconnaître la dimension « subie » de cette implication aurait été, en réalité, amputer son histoire commune avec commune avec la République. Je suis convaincu que la République se grandit chaque fois qu'elle endosse ses responsabilités, sans qu'il s'agisse nécessairement de faire acte de repentance. Il en est ainsi avec l'article 1 du projet de loi organique.

Il s'agit d'une avancée historique, et pas seulement symbolique, qui vient parachever le processus de réparation en prenant en compte et en inscrivant dans la loi cette part de l'histoire commune, dans des termes qui correspondent à la manière dont elle a été vécue par les Polynésiens. À cet égard, la sanctuarisation de la « dette nucléaire » est elle aussi une disposition de nature à sceller une relation de confiance entre la collectivité et l'État. En outre, en matière institutionnelle, le texte organique protège la stabilité de l'assemblée territoriale en corrigeant une « malfaçon pour reprendre les termes du rapporteur, par la suppression d'une règle qui aurait pu la déstabiliser en cas de mise en oeuvre. Les autres dispositions institutionnelles visent, quant à elles, à une meilleure articulation et une plus grande fluidité dans le fonctionnement des institutions. Une autre avancée concerne le contentieux des lois du pays. De fait, cette procédure révisée et la modification des délais du contrôle exercé par le Conseil d'État contribuent à sécuriser le corpus juridique local et à assurer la lisibilité des règles. C'est cela aussi, l'État de droit, et l'on ne peut que se réjouir chaque fois qu'il progresse et lorsque son fonctionnement est amélioré sur le territoire, y compris à l'échelon local. Si le transfert de la compétence est une responsabilité qui implique de veiller au strict respect de la hiérarchie des normes, il n'en demeure pas moins qu'un délai trop long pour l'entrée en vigueur des règles peut fragiliser la mise en oeuvre d'une politique publique ou rendre le droit La collectivité de Saint-Barthélemy a eu l'occasion de l'éprouver en matière pénale, certes dans une moindre mesure, certaines sanctions des infractions aux règles fixées par la collectivité n'ayant été adoptées qu'au bout de trois ans, faute d'exercice du contrôle de l'État dans un délai raisonnable. Je relève également l'encouragement à la mutualisation des compétences à l'échelon communal et la mise en oeuvre d'un principe de subsidiarité local, à l'échelle intercommunale. S'agissant d'un territoire grand comme l'Europe- on ne cessera jamais de le rappeler -, les intercommunalités peuvent être les leviers d'une planification stratégique et de développement réussie. Par ailleurs, je ne bouderai pas mon plaisir et saluerai les mesures concernant l'indivision foncière, largement issues des travaux de la délégation sénatoriale aux outre-mer, que j'ai l'honneur de présider. En Polynésie En Polynésie française, comme dans les autres territoires du Pacifique, l'enjeu réside dans l'équilibre à trouver entre la sécurisation des droits et le respect des identités locales, en particulier des pratiques sociales. Les recommandations de la délégation en matière d'indivision ont trouvé une application concrète dans la proposition de loi du député Serge Letchimy, elle-même déclinée dans le présent projet de loi ordinaire. Le texte final est très satisfaisant, mais j'ai noté la déception exprimée par notre collègue Lana Tetuanui à la suite de la suppression de l'article 14 du texte, qui prévoyait un rapport du Gouvernement au Parlement portant sur l'intelligibilité et l'accessibilité de la loi en Polynésie. Je dois le dire, si j'approuve cette suppression, fidèle à la position régulièrement affirmée par le Sénat sur les demandes de rapport, je comprends néanmoins, parallèlement, le point de vue de notre collègue. Celui-ci exprime une réalité ultramarine, à laquelle s'applique un droit qui ne lui est pas toujours adapté, quand les particularités des outre-mer n'ont pas été prises en compte au moment de la rédaction d'un texte. Je me permets donc de suggérer, à la faveur de cette disposition, que, à défaut de prise en compte originelle de ce problème, une réflexion soit conduite sur la portée des avis rendus par les collectivités lorsque celles-ci sont consultées sur les projets de textes qui leur sont ensuite applicables. Le sujet me semble concerner l'ensemble des collectivités d'outre-mer. Enfin, le texte rédigé par la commission mixte paritaire est le fruit d'un compromis respectueux du travail du Sénat, qui l'avait adopté à l'unanimité ; ses orientations ne peuvent donc que recueillir l'assentiment du groupe

Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, aucun amendement n'est recevable, sauf accord du Gouvernement ; en outre, le Sénat étant appelé à se prononcer avant l'Assemblée nationale, il statue d'abord sur les éventuels amendements, puis, par un seul vote, sur l'ensemble du texte.

je vais mettre aux voix l'ensemble du projet de loi portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire. Personne

sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant création de l'Office français de la biodiversité et de la chasse, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement, ainsi que du projet de loi organique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

effectif et direct des petites et moyennes entreprises à la commande publique, examinées au sein de son espace réservé du jeudi 13 juin 2019. Y a-t-il des observations ? ... Acte est donné de cette demande.

Monsieur le président, monsieur le rapporteur, cher Michel Laugier, mesdames, messieurs les sénateurs, il n'y a pas de démocratie sans une presse libre.

Le jour où [ ...] on verrait [ ...] la liberté de la presse s'amoindrir [ ...], ce serait en France, ce serait en Europe, ce serait dans la civilisation tout entière l'effet d'un flambeau qui s'éteint Ce flambeau, nous ne pouvons pas et nous ne le laisserons pas s'éteindre. Si nous voulons le maintenir allumé, il faut aujourd'hui raviver sa flamme si nous voulons protéger la presse, sa liberté et son pluralisme, il faut aujourd'hui moderniser sa distribution. C'est tout l'objet du projet de loi que vous examinez aujourd'hui. « loi Bichet », a souvent été qualifiée, y compris dans cet hémicycle, d'« icône de la République ». Dans le contexte tourmenté de l'après-guerre, elle avait permis de garantir l'effectivité du principe constitutionnel de pluralisme des courants de pensée et d'opinion. Comme l'a affirmé le Conseil constitutionnel dès 1984, la libre communication des pensées et des opinions ne peut être effective que si le public est à même de disposer d'un nombre suffisant de publications de tendances et de caractères différents. Cela implique que tous les journaux d'information politique et générale soient disponibles sur l'ensemble du territoire national. C'est une condition de l'effectivité de la liberté de la presse. Aujourd'hui, les objectifs de la loi Bichet demeurent garantir la pluralité de l'information et l'égalité entre les éditeurs, indépendamment de la taille de ceux-ci ou des opinions qu'ils véhiculent. les enjeux du numérique rendent cette loi encore plus nécessaire. D'une part, la diffusion numérique présente les mêmes enjeux au regard des objectifs de pluralisme ; c'est d'ailleurs pourquoi le projet qui vous est soumis prévoit l'extension des principes fondamentaux de la loi Bichet à la diffusion numérique. D'autre part, je crois profondément à l'avenir de la presse papier, à son ancrage dans nos territoires et à son utilité pour le débat démocratique. Le secteur est aujourd'hui confronté à des bouleversements importants.

Vous connaissez aussi les difficultés économiques récurrentes rencontrées par la société Presstalis, messagerie qui assure aujourd'hui la distribution de l'intégralité des quotidiens nationaux. entreprise a bénéficié d'un plan de continuation, homologué en mars 2018 par le tribunal de commerce, auquel l'État a contribué par un prêt d'un montant de 90 millions d'euros. Elle affichera cette année des fonds propres négatifs à hauteur de 400 millions d'euros. Cette situation rend donc indispensable l'adaptation de la loi Bichet. Si celle-ci est une icône de la République, elle ne doit pas en être un totem ; ce n'est qu'à condition d'être modernisée qu'elle pourra continuer à remplir les objectifs démocratiques qui lui sont assignés. Moderniser la distribution de la presse au numéro sans casser le système actuel : voilà la tâche délicate qui nous incombe. Cette tâche est délicate, parce qu'il n'est pas aisé de modifier un texte aussi ancien, aussi symbolique.

Je crois pourtant que le projet présenté par le Gouvernement parvient à résoudre cette équation, parce qu'il est le fruit d'un travail long, approfondi et mené en concertation constante avec l'ensemble du secteur. secteur. Il s'agit d'un texte équilibré et protecteur de l'intégrité de la distribution de la presse. Il permet ainsi de préserver la diversité des publications, garante de l'expression de la pluralité des opinions,

Oui, ce projet de loi préserve les principes essentiels de la loi Bichet, ce socle sur lequel notre réseau de distribution s'est construit. Il préserve le principe coopératif obligatoire, auquel est très attaché l'essentiel des acteurs de la filière,

loi préserve également le droit absolu à la distribution de l'ensemble des titres d'information politique et générale, qui resteront libres de choisir les points de vente où sont distribués leurs titres et les quantités servies. Il préserve enfin un système permettant l'accès, sur l'ensemble du territoire national, à une grande variété de publications. En effet, si la France est le pays qui propose le plus grand nombre de titres en Europe, c'est grâce à la loi de 1947, c'est grâce à la loi Bichet. Bichet. Dans sa rédaction actuelle, cette loi pose toutefois un certain nombre de difficultés, sur lesquelles les nombreux rapports et analyses menés depuis plus de dix ans nous ont éclairés. Tout d'abord, la détention majoritaire obligatoire du capital des messageries par les éditeurs place, de fait, ces derniers- à la fois clients et actionnaires -dans des situations structurelles de conflit d'intérêts. Ensuite, alors qu'ils assurent le rôle essentiel d'interface commerciale avec le client lecteur, les marchands de journaux n'ont aujourd'hui aucun contrôle sur le type de publications qu'ils reçoivent, ni sur les quantités d'exemplaires livrées. Il nous faut rendre une vraie marge de manoeuvre à ces acteurs essentiels de la filière, ainsi qu'à leurs capacités d'adaptation aux réalités du marché. Enfin, les organes de régulation de la filière disposent de prérogatives et de moyens trop limités. Sans que soit en cause la qualité du travail réalisé par les équipes du Conseil supérieur des messageries de presse, le CSMP, et de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse, à rendre sincèrement hommage à ces organismes, pour leur engagement constant au soutien de la modernisation de la filière, dans une situation souvent compliquée -, la régulation n'est pas suffisamment adaptée pour accompagner efficacement la modernisation de la filière et garantir sa pérennité. messieurs les sénateurs, vise à remédier à ces importants dysfonctionnements, sans remettre en cause les principes essentiels que j'ai précédemment rappelés. Nous proposons une vraie modernisation du cadre législatif, avec des modalités et un calendrier permettant d'accompagner la transition.

Autorité des pouvoirs d'intervention forts, en particulier en ce qui concerne l'homologation des barèmes, et en lui confiant un pouvoir de sanction dont étaient dépourvus le CSMP et l'ARDP. deuxième lieu, la fin de la détention capitalistique majoritaire des messageries par les coopératives d'éditeurs doit permettre de faire émerger de nouvelles perspectives de stratégies industrielles, pour les acteurs actuels. Elle aura également pour effet, à moyen terme, d'autoriser, le cas échéant, d'autres acteurs à proposer un service de distribution de la presse, à condition- je veux insister sur ce point soient agréés par l'Arcep sur le fondement d'un cahier des charges strict, établi par décret. Toutefois, la possibilité pour l'Arcep de délivrer des agréments à d'autres acteurs que les deux messageries actuelles ne pourra intervenir qu'après une phase de transition. En effet, le présent projet de loi autorise le Gouvernement à différer, jusqu'au 1 janvier 2023, la publication du cahier des charges définissant les conditions de l'agrément ; c'est exactement ce que nous voulons faire. le Gouvernement entend utiliser toute cette marge de manoeuvre, afin de laisser aux acteurs actuels un délai raisonnable pour s'adapter. En troisième lieu- ce point revêt une importance toute particulière dans nos territoires -, le texte prévoit de donner plus de souplesse aux marchands de journaux dans le choix des titres qu'ils distribuent, en dehors de la presse d'information politique et générale. Cet axe essentiel de modernisation doit permettre d'améliorer leur attractivité commerciale et de proposer une offre plus adaptée aux attentes des lecteurs dans nos régions, nos départements et nos communes. Les marchands de journaux y trouveront un nouveau souffle, qui ne pourra que renforcer l'attractivité d'un métier aujourd'hui affaibli par des conditions difficiles quatrième lieu- c'est tout l'enjeu d'un texte moderne, adapté à la réalité des usages de nos concitoyens -, le projet de loi étend les principes de la loi Bichet à la diffusion numérique, d'une part, en prévoyant un droit d'accès des éditeurs de titres d'information politique et générale

enfin, le projet de loi que nous présentons confie à l'Arcep la mission d'élaborer un schéma d'orientation de la distribution de la presse. Ce schéma d'orientation devra intégrer le rôle joué par les dépositaires régionaux de presse, dans une logique d'accompagnement de la transition. Ces grands axes offrent, je le crois, un cadre équilibré à l'indispensable évolution du dispositif actuel de distribution de la presse au numéro, dont la pérennité est essentielle pour l'équilibre économique de l'ensemble de la filière.

Ce projet de loi s'inscrit dans un cadre plus large : celui de la politique du Gouvernement en faveur de la presse. La directive sur le droit d'auteur, adoptée le 15 avril dernier par les institutions européennes, prévoit la création d'un droit voisin pour les éditeurs de presse et les agences de presse ; elle est déjà en cours de transposition.

Nous sommes le premier pays européen à procéder à la transposition de cette directive ; c'est la garantie, pour les éditeurs et agences de presse, de bénéficier enfin de revenus pour l'exploitation de leurs articles par les plateformes numériques. Par ailleurs, les principaux éditeurs de la presse d'information politique et générale ont présenté au ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, et à moi-même un plan de filière, afin de mieux accompagner la modernisation du secteur.

: à la distribution physique- portage, transport postal et distribution au numéro -, au pluralisme, pour les titres à faibles ressources publicitaires, mais également à la modernisation et à l'émergence de médias de proximité. aides sont essentielles à la vitalité de notre débat démocratique et à l'accès de nos concitoyens à une information fiable et diversifiée. Mesdames, messieurs les sénateurs, ensemble, c'est une nouvelle page de l'histoire de la presse écrite que nous écrivons. Ensemble, c'est l'avenir de ce secteur que nous construisons. Pour cela, nous repartirons non pas de zéro, mais des indispensables acquis de la loi Bichet. C'est tout le sens du projet de loi que vous examinez aujourd'hui.

nous ne nous arrêterons pas là ; je souhaite que nous puissions porter, auprès de la nouvelle Commission européenne, la renégociation de la directive sur le commerce électronique, qui constitue aujourd'hui, malheureusement, une entrave à notre volonté de responsabilisation des plateformes. D'autres États européens sont prêts à mener ce combat avec nous. Je veux également saluer les débats fructueux et le travail approfondi mené par la commission de la culture, de l'éducation et de la communication,

Je pense en particulier à l'amendement ayant pour objet que la commission du réseau du CSMP recueille l'avis du maire pour les décisions d'implantation des points de vente ; vous étiez très attentif à ce point, monsieur le rapporteur. Je pense aussi

D'autres amendements ont visé à clarifier le détail de la réforme et à faciliter la pleine compréhension des objectifs de celle-ci. Grâce à ces précisions, vous avez renforcé la lisibilité du texte initial, afin de lever tout risque d'ambiguïté dans l'interprétation des dispositions. Vous avez apporté des réponses aux inquiétudes de certains acteurs. Le texte ressort significativement amélioré de l'examen en commission. Mesdames, messieurs les sénateurs, au moment où je suis amené à défendre, en parallèle, quatre textes de loi devant le Parlement, je suis sensible à votre mobilisation. Vous montrez qu'il y a des causes capables de nous rassembler, de nous fédérer, des causes qui méritent que l'on dépasse nos engagements partisans. La défense du pluralisme en fait partie. La parole est à M.

Ce texte, que nous attendions depuis longtemps, réforme en profondeur l'un des piliers de notre démocratie, à savoir la loi Bichet du 2 avril 1947. Je note au passage que vous avez déposé ce texte en premier lieu sur le bureau du Sénat,

Il est rare que nous soyons appelés à réviser en profondeur une loi issue des travaux du Conseil national de la Résistance, adoptée alors que Paul Ramadier était le Président du Conseil du dernier gouvernement d'union nationale, rassemblant toutes les forces politiques issues de la Libération

En protégeant le pluralisme, c'est une condition nécessaire et essentielle du débat politique que la loi Bichet a confortée. Pour autant, pour des raisons bien connues- crise de la vente de la presse au numéro, menaces persistantes sur Presstalis -, nous sommes tous convaincus de la nécessité de faire évoluer cette loi emblématique. Vous avez hérité, monsieur le ministre, d'une situation complexe, avec de forts intérêts en jeu. Si vous avez capitalisé sur les travaux lancés par Françoise Nyssen- notamment le rapport de Marc Schwartz -, il vous est revenu de trancher et de proposer une solution, ce qui n'est jamais chose aisée, surtout dans un secteur qui déchaîne volontiers les passions. Cela doit être porté à votre crédit, de même que le pragmatisme de votre réflexion. Au moment de l'examen de la loi de finances, j'avais évoqué les quatre points qu'une réforme de la loi Bichet se devait de traiter premièrement, préserver une diffusion sur l'ensemble du territoire des titres d'information politique générale, qui est garantie par le Conseil constitutionnel ; deuxièmement, créer les conditions d'un équilibre économique durable du secteur troisièmement, redonner une place centrale aux diffuseurs de presse, les oubliés de ces dernières années ; quatrièmement, et enfin, prendre en compte l'évolution de la presse, avec la place grandissante réponse à ce programme, que j'admets ambitieux, me paraît dans l'ensemble satisfaisante. Votre réforme conserve le cadre historique de la loi Bichet, non seulement de manière formelle, mais également dans ses grands principes : la préservation d'un système spécifique et unique au monde de distribution de la presse, qui tient compte de la place éminente reconnue à la presse d'information politique et générale, et le maintien du système coopératif. Le nouveau cadre que vous nous avez proposé peut se résumer autour de trois grands principes, que vous avez évoqués à l'instant. Premier principe, la régulation serait intégralement confiée à l'Arcep il serait donc mis fin à l'autorégulation du secteur. La nouvelle autorité de régulation devrait notamment veiller à ce que les nouvelles sociétés agréées, qui assureront, à compter de 2023, la diffusion des journaux sur le territoire, agissent bien dans le respect des objectifs d'intérêt général qui sont attachés à la presse. Second principe, les diffuseurs de presse seraient enfin placés au centre du système, avec la possibilité de mener une réelle politique commerciale. À l'accès illimité au réseau, qui a contribué à l'engorgement des linéaires, succédera, une fois précisé que la presse d'information politique et générale conserve un droit absolu à être distribuée, une négociation pour déterminer l'assortiment servi dans les différents points de vente. Troisième principe, la prise en compte de la diffusion numérique de la presse, qu'elle soit le fait des kiosques numériques ou des agrégateurs. Cela rejoint pleinement les convictions fortes de la commission sur la nécessité de réguler le monde numérique. Je pense notamment à la résolution européenne sur la responsabilité partielle des hébergeurs, adoptée par le Sénat

La commission de la culture a travaillé sur ce texte de manière très ouverte, comme en témoignent les 22 amendements adoptés, issus de quatre groupes différents. En dépit des interrogations légitimes que nous pouvons entretenir sur un sujet de cette importance, nous avons travaillé selon trois axes. Tout d'abord, nous avons cherché à garantir une régulation plus efficace et plus transparente, avec l'extension des pouvoirs de l'Arcep et la possibilité pour les commissions parlementaires de saisir l'Arcep sur la question de la distribution de la presse. Ensuite, nous avons souhaité confirmer la place des diffuseurs de presse au centre du système et leur insertion dans les territoires, avec en particulier la consultation du maire de la commune concernée avant toute décision d'implantation. Enfin, la commission a estimé nécessaire de travailler à la sécurisation des conditions de diffusion, notamment à la sécurisation de l'agrément par une mention dans le cahier des charges des fonctions logistiques et financières que doivent respecter les sociétés agréées et une garantie concernant la continuité de la distribution à l'issue de la période de transition. Une fois ce cadre posé, monsieur le ministre, en saluant l'ambition et, une nouvelle fois, le pragmatisme de votre réforme, je dois vous faire part des points de vigilance, voire d'alarme, qui ont été longuement débattus par la commission. Le premier, le plus évident, est la situation de Presstalis. La réforme sur laquelle vous nous invitez à nous prononcer n'entrerait pleinement en vigueur qu'en 2023. Ce temps a été jugé nécessaire pour permettre aux acteurs existants de se préparer, ainsi qu'aux futurs candidats de réfléchir à l'opportunité d'investir le marché, ce que nous ne contestons pas. Cependant, dans le même temps, la situation de Presstalis devient critique, à tel point qu'il n'y a plus sur la table que trois solutions : un nouveau soutien massif et rapide de l'État

Je connais, monsieur le ministre, votre détermination sur ce dossier et vos propos en faveur d'un adossement. Cet état d'esprit est-il cependant partagé par vos collègues du Gouvernement ? Je pense plus particulièrement à Bercy. Très sincèrement, pouvons-nous imaginer que, d'ici à quelques mois, la presse ne soit plus distribuée en France parce qu'il y aura eu trop de tergiversations ? Tant que perdure cette attente, et malgré la qualité des équipes en place, comment Presstalis peut-il se montrer conquérant, ambitieux, et engager son renouveau sereinement ? Votre réforme de la loi Bichet fraîchement adoptée, avec son cadre ambitieux et ses principes renouvelés, trouverait à son lancement un champ de ruines, si une stratégie n'était pas rapidement adoptée et portée au plus haut niveau. Monsieur le ministre, à ce jour, et au-delà des voeux pieux, que pouvez-vous nous dire très précisément sur les discussions en cours et leurs chances de succès ? Le second sujet d'inquiétude est l'assortiment. Pour en finir avec l'accès au réseau pour tous, vous proposez de répartir la presse en trois familles. Si nous sommes pleinement rassurés sur la presse d'information politique et générale, il est aujourd'hui bien difficile de mesurer l'impact sur la diversité et le pluralisme des nouvelles règles, qui font intervenir à la fois un accord interprofessionnel et des conventions passées directement par les diffuseurs. L'amendement adopté en commission sur l'initiative de notre collègue Jean-Pierre Leleux tend à apporter une réponse que je crois pertinente, avec un « droit de présentation » pour tous les éditeurs de la presse dite « CPPAP » non retenus dans l'assortiment, ainsi que pour la presse dite « hors CPPAP Cependant, bien des inconnues subsistent. Je souhaite que notre séance soit l'occasion pour vous de nous rassurer pleinement sur cette question fondamentale, qui conditionne, dans les faits, le succès démocratique de la réforme. Monsieur le ministre, comme vous le voyez, c'est avec bienveillance, mais aussi vigilance et exigence que nous examinons aujourd'hui votre projet de loi. Avant de conclure mon propos, je voudrais dénoncer, dans les termes les plus vifs, les opérations de blocage menées par certains sur une sélection de titres détenant la qualification IPG, qui n'ont pas pu être diffusés dans les temps la semaine dernière et aujourd'hui. Nous ne pouvons que condamner avec la plus grande force cette méthode, qui, sous couvert de défendre la loi de 1947, s'en prend aux éditeurs, compromet la situation des messageries, accroît les difficultés des diffuseurs. En un mot, c'est la négation de l'esprit de la loi Bichet. J'espère, monsieur le ministre, que vous prendrez toutes les mesures pour faire cesser ce véritable scandale. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je vous remercie de votre attention, et forme le voeu que, de nos débats de ce jour, puisse sortir une nouvelle loi en mesure de conforter l'avenir de l'ensemble de la filière. La parole

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le texte que nous examinons aujourd'hui touche à un point sensible de notre système démocratique, à savoir le pluralisme et le libre accès des citoyens à des informations et des analyses diversifiées. Il concerne un maillon décisif de cette liberté démocratique : la distribution de la presse. Il s'agit en vérité d'un enjeu politique et démocratique essentiel. Il y a plus de soixante-dix ans, à la Libération, la loi Bichet, qui régit jusqu'à aujourd'hui les principes de la distribution, était adoptée, pour garantir une diffusion libre et impartiale de la presse écrite sur l'ensemble du territoire national. Après des années d'interdiction pour les uns et de collaboration pour les autres, la presse était en ruines. Elle renaissait avec la Libération, les principes de la loi Bichet visant à assurer « la liberté de la presse, son honneur et son indépendance à l'égard de l'État, des puissances d'argent et des influences étrangères ». Elle jetait les bases de trois principes fondateurs : liberté de la diffusion, impartialité de la distribution, fonctionnement coopératif et solidaire. Ces principes conservent une totale actualité. Le projet de loi récrit quasiment totalement la loi Bichet, en prétendant en conserver les principes pour la presse imprimée, et en étendre le bénéfice à la presse numérique. Une telle extension de principe est bienvenue. Toutefois, les garanties d'application exigées des grandes plateformes numériques restent extrêmement faibles et floues dans la rédaction du projet de loi. Surtout, ce texte permet-il de garantir le renouvellement des principes de la loi Bichet dans une situation où la presse est totalement bouleversée ? Nous ne le pensons pas, et nous avons les plus grandes inquiétudes sur les effets dévastateurs en termes de pluralisme de l'application d'un tel projet. Je voudrais formuler à ce propos trois grandes vous bouleversez d'abord l'organisation de la distribution en portant le coup de grâce au système coopératif, qui devait permettre de solidariser les éditeurs autour des grands principes de distribution. En vérité, les sociétés coopératives de messagerie de presse disparaissent à terme, au profit d'une libéralisation du secteur de la distribution, avec l'entrée de nouveaux acteurs sur le marché, les futures sociétés agréées prévues par le projet de loi. Vous maintenez des sociétés coopératives de groupage de presse, que les éditeurs pourront créer, mais pour soumettre leur distribution à des sociétés agréées concurrentes. Nous allons donc entrer dans une concurrence exacerbée des éditeurs et des sociétés agréées. Vous justifiez Vous justifiez ce basculement par la crise actuelle, très réelle, du secteur de la presse et de la distribution, mais vous n'en traitez pas la cause ; au contraire, vous soignez le mal par le mal. Dans une situation de baisse marquée des ventes, les gouvernements ont laissé perdurer, malgré les alertes,

Oui, une grande réforme était nécessaire pour faire revivre les principes de la loi Bichet, avec la reconstitution d'un grand opérateur unique, coopératif, doté de moyens et d'acteurs publics nouveaux, comme La Poste, et et une stratégie publique renouvelée en matière de numérique face aux plateformes qui pillent le secteur à sens unique. Toutefois, vous choisissez la voie inverse, celle de la concurrence renforcée, avec tous les risques qu'elle fait courir au pluralisme et à de très nombreux titres, aujourd'hui économiquement fragiles, mais indispensables à nos libertés démocratiques. Devant les risques encourus, vous affirmez maintenir pour chaque titre le droit à être distribué. Vous l'inscrivez dans la loi pour la presse d'information politique et générale, et vous comprendrez combien nous sommes attachés à une telle disposition. Mais vous différenciez ensuite ce droit pour les différentes catégories de presse ; c'est un engrenage dangereux.

de principe inscrite dans la loi d'une distribution non discriminatoire. Qui garantira que le système n'aboutit pas à une situation inverse aux principes énoncés ? Vous instituez un nouveau régulateur, l'Arcep, auquel vous confiez tous les pouvoirs de régulation. Mais en noyant la régulation de la presse, sujet éminemment politique, dans une autorité de régulation dominée par les enjeux de concurrence des grands acteurs du numérique et de la logistique, vous prenez, là encore, le risque d'aggraver les logiques d'écrémage du pluralisme. C'est notre second point d'inquiétude.

À la concentration dans les mains de ces puissances d'argent de la propriété d'une part sans cesse grandissante des médias d'information, vous ajoutez le risque d'une mainmise de ces puissances sur la distribution, c'est-à-dire d'un droit de vie ou de mort sur plusieurs dizaines de titres de presse. Car la concurrence que vous ouvrez aboutira tôt ou tard à une concentration accrue et à la reconstitution de monopoles privés sur la distribution. Voilà pourquoi, monsieur le ministre,

mes chers collègues, le projet de loi dont nous discutons aujourd'hui était annoncé depuis longtemps. Le rapport Schwartz, rendu en juin 2018, avait donné au Gouvernement des orientations pour sa rédaction. On peut cependant regretter le calendrier législatif,

un compromis. Ces délais sont trop courts pour réformer un texte qui est l'un des joyaux législatifs issus de l'oeuvre fondatrice du CNR, une loi « icône », comme je l'avais déjà qualifiée en 2011. Elle découle directement d'une exigence constitutionnelle, posée à l'article XI de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui garantit la libre communication des opinions. Ainsi, la loi Bichet avait permis d'assurer des principes qui restent d'actualité : la liberté de la diffusion de la presse imprimée et l'égalité de traitement entre tous les titres, quel que soit leur poids

Bien sûr, depuis 1947, l'écosystème de la presse, de la production d'informations, des supports, de l'édition, de la communication au public, de son acheminement et de sa vente a été fortement bouleversé. Il se vend beaucoup moins de journaux papier, le nombre de quotidiens a baissé et la vente s'est effondrée de 56 % entre 2007 et 2017, sans qu'il soit possible de dire si nous avons atteint un palier. la diffusion individuelle du est majoritairement numérique. C'est un mouvement qui touche l'ensemble de la presse quotidienne nationale et qui commence à se développer fortement pour les autres titres. Par souci de valoriser la presse d'information politique et générale sur internet,

qui concerne la diffusion de la presse papier, qui est le coeur du texte, je ne partage pas l'optimisme de M. le rapporteur quand il affirme que le projet de loi tient à conserver les principes de la distribution de la presse tels qu'ils ont été sanctuarisés par la loi Bichet jusqu'à présent.

la messagerie transporte l'ensemble de notre presse quotidienne nationale et joue un rôle capital dans le système actuel. Le projet de loi prévoit l'arrivée, avant 2023, et non à partir de cette date, d'un nouvel acteur. Pourtant, la société est en pleine restructuration. Un plan de sauvetage a été adopté en 2018 et mis en place depuis lors. Alors que Presstalis remonte la pente depuis deux ans, avec un plan de redressement et de sauvegarde de l'emploi, déjà fortement réduit ces dernières années, notamment en planifiant un volet de développement commercial nécessaire à sa survie, alors que les clients commencent à revenir, cette loi prévoit l'arrivée d'un nouvel entrant- ou de plusieurs -sur le marché de la distribution dès son adoption. Cette annonce a déjà eu pour effet de geler l'effort de Presstalis et d'arrêter net tout nouveau contrat : les éventuels clients - c'est logique ! - préfèrent attendre de voir quel opérateur tirera son épingle du jeu suscité par la nouvelle législation. La société ne peut donc poursuivre son développement avec une pareille incertitude. La courbe ascendante est stoppée net, d'autant que, cette semaine, la Cour des comptes a émis des doutes sur la mise à disposition de crédits pour le Fonds stratégique pour le développement de la presse, dont le montant va baisser, poussant le contrôleur budgétaire à poser ouvertement la question de savoir si les crédits ne manqueront pas pour la transformation stratégique du secteur.

Il s'agit simplement d'une garantie de stabilité pour ces entreprises et leurs personnels. Nous nous satisfaisons

des barèmes, afin que l'ensemble des éditeurs sache à quoi s'attendre en rentrant dans une société de distribution de presse. Sur ce point, je suis heureux que la commission nous ait suivis. M. le ministre

L'agrémentation des sociétés qui effectueront la distribution de la presse permettra de contrôler en amont les motivations d'un opérateur et sa capacité à assurer la distribution, en termes économiques, mais aussi pour ce qui concerne le maillage du territoire,

à savoir les kiosquiers. La vente au numéro ne cesse de s'éroder, et la disparition des marchands de journaux, de nous émouvoir. Entre 2011 et 2017, quelque 5 300 points de vente ont été fermés, soit une baisse de 19 %. La filière estime que le réseau devrait se réduire à 21 000 points de vente en 2020,

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le texte que nous examinons aujourd'hui est d'une importance capitale pour la vitalité de notre presse écrite et, donc, de notre démocratie. Bien des choses ont été dites sur le quatrième pouvoir, que les médias forment aux côtés du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif et de l'autorité judiciaire. À l'époque où il était ministre délégué de la communication, André Santini considérait déjà que les médias avaient remplacé le pouvoir législatif dans sa fonction de mise en scène du débat public. Leur utilité démocratique justifie qu'une protection légale, conventionnelle et constitutionnelle leur soit accordée, comme le prévoient aujourd'hui le droit français et le droit européen. Pour autant, la situation actuelle de la presse écrite nous rappelle qu'il s'agit d'un pouvoir fragile, exposé aux mutations technologiques, aux appétits des grands groupes et aux tentatives d'instrumentalisation politique. D'ailleurs, lorsque la loi Bichet avait été adoptée en 1947, l'âge d'or de la presse écrite française semblait déjà derrière elle. Celle-ci subissait la concurrence de la radio, avant celle de la télévision, qualifiée de « bourrage de crâne » par Albert Londres, et elle était accusée de corruption au moment de l'affaire des emprunts. Le secteur de la distribution de la presse n'est pas un secteur économique comme les autres : il figure au rang des « monopoles naturels », ce qui justifie l'intervention de l'État. le Conseil national de la Résistance avait d'ailleurs favorisé le démantèlement du monopole du groupe Hachette, celui-ci ayant été établi grâce à son entregent politique sous le Second Empire et à sa bonne entente avec les dirigeants des chemins de fer. Sans le régime de distribution coopératif, particulièrement avantageux, de la loi Bichet et l'existence de tarifs postaux préférentiels, dont la création est plus ancienne, la reconfiguration du paysage médiatique français aurait été plus radicale et peut-être plus exposée aux assauts de « moguls » étrangers, comme ceux de Rupert Murdoch contre la presse anglo-saxonne. Si un regard extérieur est toujours instructif, nous sommes tous convaincus ici de la nécessité de maintenir les conditions d'existence d'une presse française indépendante, ce qui passe aujourd'hui par une adaptation du régime de sa distribution aux nouvelles circonstances de notre époque. En effet, dans l'énorme masse des analyses et commentaires diffusés en continu à la radio, à la télévision et sur les réseaux sociaux, la presse écrite fait désormais office de référence. Les grandes plumes et les éditorialistes continuent d'influencer la polarisation des débats dans toutes les strates médiatiques. Attachés comme nous le sommes à l'état de droit, nous reconnaissons à la presse la qualité de respecter des principes déontologiques forts, qui ébranlent les rédactions lorsqu'ils sont bafoués, montre aujourd'hui l'affaire Claas Relotius au, sans oublier les vertus de l'engagement de la responsabilité des journalistes en leur nom propre, alors que, à l'heure du tout numérique, la tentation de l'anonymat et du pseudonyme permet toutes les dérives et toutes les infox. C'est pourquoi nous sommes particulièrement sensibles à la triple crise du système de distribution auquel nous assistons : crise structurelle, liée à la migration numérique et à la marginalisation du papier ; crise économique de l'acteur incontournable qu'est Presstalis ; enfin, crise de la gouvernance du régime de distribution de la presse. Au regard de l'effondrement des ventes du papier et de la multitude des intérêts contraires en présence, nous considérons que le texte examiné permet des équilibres très satisfaisants. des équilibres très satisfaisants. Il offre de solides garanties pour préserver le pluralisme, tout en réorganisant le niveau 2 de la distribution, afin d'en renforcer la viabilité économique. Ni la liberté de la presse ni le principe coopératif de la distribution ne sont remis en cause, et la création d'un nouvel échelon de sociétés agréées contractant avec les sociétés coopératives permettra d'accompagner la modernisation des systèmes d'information entre éditeurs et points de vente. C'est le résultat du travail rigoureux et de l'esprit constructif du Gouvernement et de M. le rapporteur, Michel Laugier, que je remercie. Les amendements que nous proposons visent à s'appuyer sur cet équilibre pour renforcer les garanties apportées chacun des acteurs, dans le sens du pluralisme et de la préservation d'un maillage territorial satisfaisant. Nous serons particulièrement vigilants au sort réservé aux kiosquiers et aux maisons de la presse répartis sur l'ensemble de notre territoire : ils sont les héritiers des bibliothèques de gare, qui ont pris une part importante dans l'instruction publique de notre pays. Quant au nouveau système de gouvernance proposé, vous connaissez la position de méfiance du groupe RDSE à l'égard des autorités administratives indépendantes. Toutefois, les deux instances existantes ayant échoué à faire leurs preuves, le transfert de compétences à l'Arcep nous semble relever du pragmatisme, à condition de la doter d'un pouvoir de sanction efficace ; nous y reviendrons.

Monsieur le ministre, vous le savez : la presse écrite ne disparaît pas ; elle se numérise. Au sein des rédactions, les services se réorganisent. Il convient d'accompagner cette mutation par l'instauration d'une protection du pluralisme en ligne, équivalente à celle qui protège la presse papier. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont une nouvelle courroie de distribution de la presse ; or ses règles de fonctionnement échappent à l'État, au risque de fausser le jeu démocratique, sous l'influence de puissances étrangères ou d'intérêts catégoriels. Osons aller au-devant d'une lente modification des règles européennes ; il y va de l'avenir de notre démocratie ! Nous voterons certainement ce texte.

Presstalis, principal acteur du secteur, qui distribue l'intégralité des quotidiens, présente à ce jour 400 millions d'euros de fonds négatifs. Or, avec une distribution de la presse en grande difficulté, c'est le pluralisme des opinions qui risque de chanceler. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, qui est pour beaucoup imputable au totalitarisme et au populisme, la loi Bichet rappelait le principe essentiel de la libre distribution de la presse, principe confirmé par le Conseil constitutionnel : la libre communication des pensées et des opinions exige que le public dispose d'un nombre suffisant de publications de tendances et de caractères différents. La distribution de la presse au numéro doit ainsi concourir à ce que soit atteint l'objectif à valeur constitutionnelle du pluralisme. La loi Bichet a contribué à la réalisation de cet objectif : le Conseil d'État indique que quelque 4 400 titres sont aujourd'hui distribués en France, contre 2 500 au Royaume-Uni et 1 en Allemagne. Cette réussite a néanmoins un coût, notre système prévoyant une large couverture du territoire et un nombre important de publications. Ce coût s'est trouvé aggravé par la réduction structurelle de la vente de presse papier au numéro. En dix ans, le volume de cette vente a fondu de moitié. Un tiers des points de vente ont disparu- chaque année, ce sont 1 000 points de vente qui ferment. Aussi est-il nécessaire de réformer le cadre de la distribution de la presse au numéro en France, afin de l'adapter au changement de la société et afin de renforcer l'efficacité économique du secteur. avait permis de mettre en lumière les difficultés du système actuel. La gouvernance doit évoluer, et l'efficacité économique revenir au centre de l'activité. L'objet du projet de loi que nous examinons est de réformer le secteur en douceur, si je puis dire. Il est ainsi proposé d'ouvrir la distribution de la presse au numéro à la concurrence, de manière progressive et encadrée. Le groupe Les Indépendants - République et Territoires est convaincu qu'une concurrence loyale favorisera utilement les gains d'efficacité économique et participera à l'assainissement du secteur. La mise en concurrence est selon nous nécessaire et utile ; mais cette concurrence doit être encadrée. Un tel encadrement est nécessaire pour que la concurrence soit loyale, mais aussi afin de garantir la préservation du pluralisme des opinions, si essentiel à la vie démocratique. Le projet de loi prévoit que l'on passe de deux régulateurs à un seul. Cette unification nous semble être une mesure de bon sens. Néanmoins, le choix de confier la régulation à l'Arcep a soulevé certaines critiques. Cette autorité saura-t-elle aller au-delà d'une régulation purement économique ? L'avenir nous le dira ; il appartiendra à l'Arcep de faire ses preuves. Quoi qu'il en soit, nous nous félicitons que notre commission ait veillé, tout en augmentant les compétences de l'Arcep, à rendre leur exercice plus transparent- cette évocation du travail de la commission pour féliciter notre rapporteur, Michel Laugier, de la qualité du travail effectué et du professionnalisme dont il a fait preuve tout au long de l'examen Afin de redynamiser le secteur, il est prévu de donner davantage de souplesse aux quelque 24 000 acteurs qui sont en première ligne en matière de vente de presse au numéro : les diffuseurs de presse. Nous sommes convaincus que les points de vente sont les mieux à même de connaître les attentes de leurs clients. Ils doivent être en mesure de mettre en avant les titres qui y correspondent.

Nous avons commencé à agir, avec la création du droit voisin de la presse, afin que les acteurs du numérique cessent d'exploiter les contenus des agences de presse et des éditeurs de presse sans autorisation ni rémunération. outre le sujet de la rémunération, le fait que les plateformes d'agrégation de contenus orientent sensiblement l'opinion publique, en sélectionnant les articles qu'elles présentent aux usagers. Les habitudes de consommation de nos concitoyens évoluent de plus en plus vers le numérique, au détriment de l'écrit. Il est par conséquent primordial que les usagers de la presse numérique puissent savoir sur quels mécanismes repose la présentation de l'information qui leur est Nous sommes favorables à la réglementation instituée par le texte, qui astreint les opérateurs numériques à respecter le pluralisme et les soumet à des obligations explicites de transparence.

Je constate enfin- avec regret, mais sans surprise -que la CGT a décidé d'empêcher la parution des quotidiens le jour même où le Sénat examine le projet de loi portant réforme de la vente en kiosque, qui est destiné à sauver Peut-on dire chose plus absurde, à tous ceux qui continuent à lire le journal papier, que : « Pour le défendre, nous vidons les kiosques aujourd'hui et vous forçons à vous rabattre sur la version web de votre quotidien »

que je veux la presse dans toute sa liberté », déclarait Victor Hugo devant l'Assemblée nationale législative, le 9 juillet 1850. Près d'un siècle et demi plus tard, la question de la sauvegarde du pluralisme de la presse se pose une nouvelle fois à nous, avec une acuité toute particulière.

C'est pourquoi cette réforme apparaît, d'une part, pleinement nécessaire, et, d'autre part, pertinente quant aux enjeux qu'elle a vocation à traiter. Ce projet de loi nous semble constituer une réponse pragmatique à la crise que traverse la distribution de la presse. Nous ne reviendrons pas sur le détail de la situation très précaire de Presstalis, déjà évoquée en commission,

Assurément, la forme coopérative est celle qui, depuis l'origine, permet de garantir l'équité de distribution entre les éditeurs et d'éviter toute situation d'abus de position dominante. En cela, l'article 1 permet de préserver le caractère singulier du système de distribution de presse français. De plus, le recentrage de la régulation du système autour d'une autorité unique, l'Arcep, et l'élargissement des compétences de celle-ci, vont incontestablement dans le sens d'une plus grande efficacité : efficacité en matière de régulation, puisque l'Arcep agréera les sociétés de distribution et disposera d'un pouvoir de sanction à l'encontre des différents acteurs

ensuite seulement, éventuellement, des titres de presse papier. Or légiférer sur ces agrégateurs, c'est précisément oeuvrer pour une meilleure protection des jeunes publics, souvent plus vulnérables que les autres. À cet égard, le texte vise à renforcer la responsabilité des acteurs majeurs d'internet, à savoir les agrégateurs, qu'il s'agisse d'améliorer l'information des internautes en matière d'utilisation de leurs données personnelles lesdits acteurs à rendre publics les critères qu'ils prennent en compte pour agréger les titres de presse. Bien sûr, nous encourageons ces évolutions. Mais il est difficile de ne pas poser la question de leur efficience. En un mot : les agrégateurs de presse vont-ils vraiment jouer le jeu ? Par ailleurs, s'agissant des kiosques numériques, qui posent moins de difficultés, nous considérons, nous aussi, qu'il revient au législateur d'inscrire dans la loi l'obligation pour ces sites d'accueillir la presse d'information politique et générale sur demande.

D'ailleurs, le choix du Gouvernement d'inscrire la réforme dans le cadre même de la loi Bichet, plutôt que dans un nouveau texte, est une décision particulièrement bienvenue d'un

façon, le texte prône la continuité, la neutralité et l'efficacité économique de la distribution de la presse, ainsi qu'une bonne couverture du réseau des points de vente. Ces principes doivent être et demeurer au coeur de la loi.

; il a fait preuve d'une grande clarté sur un sujet pourtant complexe, montrant par là qu'il le possède bien, de façon toute professionnelle. Comme le remarquait Jean-Paul Sartre, « on croit que le droit à la liberté de la presse, c'est un droit du journaliste. Mais pas du tout, c'est un droit du lecteur du journal ». Or le projet de loi que nous soumet aujourd'hui le Gouvernement tend précisément vers un juste équilibre entre les intérêts des acteurs de la distribution de la presse et ceux, tout aussi essentiels, des lecteurs.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme le Conseil constitutionnel a eu l'occasion de l'exprimer solennellement le 11 octobre 1984 lors de l'examen de la loi visant à limiter la concentration des entreprises de presse, le pluralisme n'est effectif que « si le si le public est à même de disposer d'un nombre suffisant de publications de tendances et de caractères différents ». Si cette affirmation nous semble aujourd'hui

Auparavant, et depuis 1789, la distribution de la presse était soumise à un monopole postal impliquant de fait un contrôle étatique et une censure préalables.

La loi Bichet visait- on le sait -à tourner définitivement la page de la sombre période qui avait précédé, où l'occupant nazi avait réquisitionné les messageries pour s'assurer un contrôle total de la presse.

dégradation de la situation économique des Messageries françaises de presse, qui avaient été instaurées en août 1945 par le Gouvernement provisoire de la République française, situation qui, au passage, n'est pas sans rappeler nos inquiétudes actuelles quant quant à la pérennité économique de la principale coopérative de distribution de la presse dans notre pays. Rappelons aussi que, à l'époque où la loi Bichet fut votée, la presse écrite était essentiellement une presse d'information et d'opinion de périodicité quotidienne : 180 quotidiens, en 1946, contre à peine 72 aujourd'hui, chiffre au demeurant très généreux,

celle de l'abondante prolifération de la presse magazine spécialisée, notamment durant les années 1970 et 1980, puis celle, plus récemment, de l'information en ligne et des réseaux sociaux, qui divulguent gratuitement des nouvelles dont il est de plus en plus rare qu'elles soient produites par des journalistes professionnels. des points de vente s'accélère, et la société Presstalis est aujourd'hui lourdement lestée de 400 millions d'euros de fonds propres négatifs. Oui, monsieur le ministre, vous avez raison de dire, concernant la réforme de la loi Bichet, qu'il faut « la moderniser sans la casser ». Le texte qui nous est présenté aujourd'hui, sous des apparences parfois complexes et même très techniques, a la grande qualité, au travers de ses compromis et ses jeux subtils d'équilibre, de respecter ce juste postulat. Il respecte notamment certains fonctionnements qui ont fait leurs preuves, tout en prenant en compte les attentes des principaux acteurs de la filière, à savoir les marchands de journaux, et les évolutions techniques autant que technologiques.

terme. Cela permet de continuer à associer les éditeurs au fonctionnement des messageries de presse, tout en offrant désormais la possibilité d'ouvrir leur capital à d'autres acteurs de la distribution.

politique et générale, et les titres CPPAP, c'est-à-dire les titres reconnus par la commission paritaire des publications et agences de presse, ils pourront, des accords interprofessionnels, choisir ce qu'ils souhaitent vendre parmi les autres titres de la presse magazine. Ils pourront ainsi adapter leur offre et se montrer plus pertinents au regard des attentes effectives de leurs clients. Cette possibilité de choix contribuera à sauver le maillage actuel des marchands de journaux, voire à le revitaliser. Le fait, par ailleurs, de confier la gestion des négociations de distribution à l'Arcep simplifie la régulation du secteur, en supprimant les deux actuelles autorités en charge de celle-ci, le CSMP et l'ARDP, qui étaient trop souvent, il faut le dire, juges et dire, juges et parties dans les arbitrages. Les compétences de l'Arcep en matière de régulation du secteur postal pourraient être très utiles s'agissant de la distribution de la presse, de même que l'ouverture offrira sur le monde des réseaux de communications, désormais essentiels à la circulation de l'information. Qu'en est-il, d'ailleurs, d'internet et de la presse écrite ? Il est précisément prévu, dans ce texte, plusieurs changements de taille. Les kiosques numériques auront notamment l'obligation d'intégrer tous les titres IPG, dans les mêmes conditions que dans l'univers physique. Autre innovation portée par ce texte : la « responsabilisation » des agrégateurs d'information, Google News, Apple News, MSN, Yahoo ! et tant d'autres, qui seront soumis à une obligation de transparence,

est en grande difficulté ; sa messagerie Presstalis est au bord du redressement judiciaire, et, avec elle, à terme, des milliers d'emplois sont menacés. Quel avenir, alors, pour la presse ? Qu'elle soit quotidienne, régionale ou magazine, c'est la grande question qui se pose à nous aujourd'hui. qui se pose à nous aujourd'hui. Internet, pour elle, a été un choc ; il l'est toujours, après plusieurs années. Son avènement a mis les journaux en difficulté et a poussé les groupes à se restructurer.

au Sénat. Cette reconnaissance est à la hauteur du travail mené par la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, sous la présidence de Catherine Morin-Desailly, et de l'investissement sans faille de notre rapporteur Michel Laugier- je tiens à les remercier, l'un et l'autre, de la grande qualité des travaux menés. Le défi à relever est de taille. En effet, nous ne vivons pas uniquement une crise de la distribution, mais aussi une profonde mutation de la presse dans notre pays. étaient tenues les sociétés de distribution d'avoir leur capital majoritairement détenu par les coopératives d'éditeurs. Ces dernières pourront ainsi contracter avec des sociétés agréées, suivant un cahier des charges précis.

D'autres interrogations demeurent sur le service rendu par ces nouveaux acteurs, et, en particulier, sur l'incidence d'une telle ouverture du marché sur le droit à l'information. À cet égard, nous avons proposé un amendement visant à garantir que les différents points de vente d'un territoire soient desservis de manière non discriminatoire. Les marchands de journaux auront par ailleurs une plus grande liberté dans la gestion de leurs stocks, compte tenu du nombre croissant de leurs invendus.

de sanction. L'Arcep aura également pour mission d'agréer les nouveaux acteurs souhaitant proposer un service de distribution de presse. Nous souhaitons toutefois insister sur la nécessité d'accompagner le régulateur dans sa nouvelle mission. Comme l'a rappelé M. Sébastien Soriano

numérique. Vous l'aurez compris, monsieur le ministre, nous ne partageons pas la vision apocalyptique d'une presse condamnée par internet, incapable de survivre sans le soutien de l'État. Nous pensons que des possibles s'offrent à elle, que des initiatives peuvent être prises. Selon la théorie de l'économiste Israël Kirzner, l'entrepreneur est celui qui saisit les opportunités

Cependant, il faut bien admettre que nous accédons désormais de moins en moins à l'information en parcourant des yeux les linéaires d'un diffuseur, et de plus en plus par voie numérique. Or je m'interroge sur la possibilité de coexistence entre un monde physique, égalitaire et régulé et un monde, de plus en plus dominant, obéissant obéissant à une logique exactement inverse, dérégulé et inégalitaire. Quand je me connecte, des algorithmes sophistiqués cherchent à capter mon attention en me présentant des contenus d'information supposés m'intéresser. Dès lors, il n'y a plus de débat, plus d'échange, plus de surprise : ce que les psychologues appellent le « biais de confirmation » joue pleinement et m'enserre dans mes certitudes. Je ne parle pas ici de quelques sites isolés, mais des fondements mêmes de l'économie de l'internet, désormais dominante, qui déferle sur la presse, mais aussi sur la musique, l'audiovisuel, le cinéma et l'ensemble des secteurs de la culture. Face à ce défi, monsieur le ministre, je reconnais que votre texte a le mérite d'essayer de faire bouger les lignes aussi loin que possible. En particulier, vous demandez aux plateformes de fournir à l'internaute « une information claire, loyale et transparente sur l'utilisation de ses données personnelles dans le cadre de la mise en avant de ces contenus ». C'est déjà beaucoup, car vous faites effectivement le lien entre l'information collectée sur l'internaute et celle qui lui est proposée. Mais

Vous le savez, le Sénat, grâce à la proposition de loi de notre collègue David Assouline, a été à l'initiative d'une transposition anticipée des dispositions de la directive Droit d'auteur relatives au droit voisin des éditeurs de presse.

de l'exercice. Mais si nous avons été capables d'être fer-de-lance sur les droits d'auteur et les droits voisins, nous pouvons l'être aussi sur la révision et la réouverture de la directive e-commerce. Disons-le, plaider

Bonhomme, sur l'article. On ne peut évidemment que souscrire à l'ambition générale affichée à l'article 1 : préserver le pluralisme et la diversité de l'offre de presse en veillant à garantir l'égalité de traitement entre éditeurs et en leur donnant la capacité d'accéder librement un large réseau de distribution.

Libre pour sa nouvelle imprimerie, dont le coût total oscillerait autour de 6 millions d'euros. Or cette subvention aurait été accordée malgré l'avis négatif de la direction générale des médias et des industries culturelles, souhaite exprimer mon étonnement devant une telle subvention, lorsque l'on sait que les règles du Fonds stratégique pour le développement de la presse, le FSDP, prévoient explicitement que le montant de l'aide susceptible d'être accordée à un projet éligible

En 2018, le montant du FSDP s'est élevé officiellement à 27 millions d'euros. Mais, au détour d'une belle acrobatie comptable, la loi de finances a « mis en réserve » 9 millions d'euros ... Autrement dit, seuls 18 millions d'euros ont effectivement pu être distribués en 2018. Ultime détournement de la finalité du fonds,

Résultat, il ne restait plus que 9 millions d'euros de subventions disponibles pour toute l'année. L'aide accordée à Midi Libre atteint ... 38 % de cette somme, dépassant largement le plafond ! Monsieur le ministre, j'espère que vous pourrez nous éclairer sur les conditions dans lesquelles ces aides ont été obtenues.

les ventes ont chuté de 56 %. Quasiment sur la même période, 5 300 points de vente ont été fermés, soit une baisse de près de 20 %. Au-delà de cet état des lieux, la tendance devrait se poursuivre à moyen terme, suscitant des inquiétudes, autant chez les éditeurs de presse que chez les distributeurs. Le Gouvernement a fait le choix de réformer la loi

la traduction concrète de trois principes-clefs : la liberté de diffusion, l'impartialité dans la distribution des journaux et la solidarité coopérative entre les journaux. Ces derniers concourent eux-mêmes au respect et à l'application d'un « méta-principe », ultérieurement d'ailleurs consacré par le Conseil constitutionnel en tant qu'objectif à valeur constitutionnelle : le pluralisme des quotidiens d'information politique et générale. Sans oublier les autres titres de presse,

En d'autres termes, les réformes substantielles affectant l'environnement économique de la distribution de la presse qui sont contenues dans ce projet de loi doivent veiller à ne pas écorner les principes philosophiques et constitutionnels qui fondent notre identité démocratique. Un savant démocratique. Un savant équilibre est donc à préserver entre recherche d'une amélioration de la situation économique des acteurs de la filière presse et conformité à nos principes démocratiques. à nos principes démocratiques. Or cette conformité passe également par une diffusion des journaux et publications autres que la presse d'information politique et générale la plus équilibrée possible sur l'ensemble du territoire. Car comment pourrait-on parler de démocratie

les principes de solidarité dans la distribution. Comme je l'ai souligné dans mon intervention liminaire, nous sommes extrêmement inquiets quant à l'avenir de ces principes de solidarité.

de cet amendement proposent d'inclure dans le système de péréquation et de prise en charge des frais les entreprises de presse à vocation nationale, qui assureraient elles-mêmes Actuellement, la seule presse à assurer sa propre diffusion sans recourir au groupage est la presse régionale. Toutes les autres familles de presse recourent aux messageries pour mutualiser les coûts, et cela ne devrait pas changer dans le futur. L'adoption d'un tel amendement n'aurait donc pas d'effet. Au demeurant, il n'existe pas de définition de la presse à vocation nationale. La commission émet

le système coopératif était maintenu. Mais maintenir le système coopératif de groupage de presse et maintenir le système coopératif de distribution, ce n'est pas pareil ! En effet, nous aurons des sociétés coopératives de groupage de presse qui délègueront la distribution à des sociétés agréées.

seront qualifiées ou non comme telles, elles garderont ou non la main sur les conditions de diffusion, notamment la quantité. En outre, l'élévation de cette définition au niveau légal rend les possibilités de recours plus difficiles en cas de difficulté. L'objet de l'amendement est de souligner les risques liés à l'inscription dans la loi du critère jurisprudentiel d'une publication devant contenir des commentaires ou analyses de nature à « éclairer le jugement Ce critère, s'il est aujourd'hui peu remis en cause, pose question du fait de sa subjectivité. N'y a-t-il pas un risque pour la commission à qui reviendra la charge de la qualification, le juge en cas de recours, d'émettre un jugement de valeur sur le travail journalistique accompli ? C'est pourquoi nous proposons de le remplacer par un autre critère, objectif celui-ci : l'existence d'une charte déontologique. Cette obligation s'impose aux rédactions depuis la loi du Cette existence permettrait de s'assurer du sérieux des contenus proposés, en respect de la charte, sans avoir à émettre de jugement de valeur de ces contenus pour le citoyen. Cette disposition est donc plus protectrice des journalistes, tout en s'inscrivant en cohérence avec les évolutions législatives récentes. Elle vise à faire en sorte que l'argument de faible éclairage du citoyen ne puisse jamais être utilisé contre un titre titre de presse IPG qui serait devenu dérangeant pour le pouvoir, quand la composition de la commission chargée de la qualification n'est pas définie dans la loi. Il s'agit donc d'amorcer une réflexion qui devrait, selon nous, se poursuivre à l'Assemblée nationale. Quel est commission ? Cet amendement vise à remplacer un critère de définition de la presse IPG tendant à éclairer le jugement des citoyens par le respect d'une charte déontologique. Le projet de loi a élevé au rang législatif la définition de la presse et de l'information de politique générale, jusque-là contenue dans l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques. Les auteurs du présent amendement proposent de modifier la définition. cela risque de fragiliser les titres actuellement en IPG et toute la jurisprudence. D'autre part, l'obligation de disposer d'une charte déontologique est déjà inscrite dans la loi Bloche. Il faudrait d'ailleurs en assurer une meilleure effectivité.

Dans son avis, le Conseil d'État a considéré qu'il s'agissait d'une disposition de nature réglementaire et proposé le renvoi à un décret. Il est vrai que c'est souvent le cas dans bien des domaines. Pour autant, s'agissant de la presse d'information politique et générale, et de l'importance de cette commission en faveur de la préservation du pluralisme, il nous paraît absolument nécessaire de prendre des précautions législatives, afin que la composition de cette commission ne puisse être modifiée dans un sens ou dans un autre, pour permettre à tel ou tel gouvernement de sanctionner un organe de presse qui serait trop critique. Il nous revient d'anticiper tous les scénarii possibles, dès lors que la loi dispose pour l'avenir. Dans ce cas précis, il aurait peut-être même été justifié de prévoir que la composition soit fixée dans la loi : cela existe dans d'autres domaines, comme pour la Commission de déontologie de la fonction publique dont il est aujourd'hui beaucoup question. Cet amendement tend également à clarifier les voies de recours,

Le présent amendement vise à inscrire l'apport de la presse étrangère dans le pluralisme nécessaire à la vie démocratique française. Faut-il rappeler que la Résistance s'est organisée depuis l'étranger et que certains médias étrangers ont eu un rôle dans la libération de notre pays ? Sans le soutien de la BBC, l'appel du 18 juin aurait probablement trouvé moins d'écho Actuellement, on compterait environ 1 400 références de presse étrangère, contre près de 4 000 pour la presse coopérative, pour un chiffre d'affaires total de 46 millions d'euros.

On imagine que les points de vente auraient donc intérêt à moins la diffuser. Comme cela l'a été mentionné dans la discussion générale, nous considérons que ce regard extérieur est très utile au pluralisme et qu'une plus faible diffusion sur notre sol affaiblirait la qualité du débat public. Contrairement aux critiques de certains acteurs de la presse contre notre amendement, celui-ci ne vise pas du tout à supprimer le régime actuel de distribution de la presse étrangère en France, qui est dérogatoire. Il ne tend pas non plus à permettre à des titres voulant contourner la qualification IPG de se localiser à l'étranger pour être mieux diffusés. Il s'agit seulement de protéger la presse IPG étrangère de la même manière que la presse IPG nationale, afin, notamment, que les points de vente ne puissent s'opposer à leur En réalité, et nous attendons que le ministre le confirme, la CPPAP opère déjà une distinction entre les titres étrangers selon qu'il s'agisse de presse IPG ou autres. Cet amendement ne nous semble pas remettre en question cette façon de faire ; et si tel était le cas, nous serions prêts à le rectifier dans le sens du droit constant. En tout état de cause, il nous paraît essentiel de rappeler que la presse étrangère doit être protégée sur notre sol au même titre que la presse nationale, afin de ne pas nourrir un isolement médiatique français. Quel est l'avis de la commission ? Cet amendement vise à instaurer une égalité de traitement entre la presse étrangère et la presse française. partent d'une idée très louable, chère Françoise Laborde, mais elles appellent quelques clarifications. La presse étrangère distribuée par les messageries en France ne fait pas partie des coopératives d'éditeurs, mais représente une activité spécifique « import pour les distributeurs. Les journaux sont cependant placés dans les mêmes catégories que la presse française : IPG, CPPAP. Cette activité est soumise à une tarification qui lui est propre et qui ne dépend donc pas aujourd'hui des barèmes votés par les coopératives. Elle représente en 2017 quelque 1 400 références, pour un chiffre d'affaires total de 46 millions d'euros, avec un taux d'invendus très important de 74 %, contre 49 % pour la presse coopérative. La réforme que nous examinons ne devrait rien changer quant au traitement de la presse étrangère, qui constituera toujours une activité spécifique pour les sociétés de distribution. Les titres bénéficieront des mêmes droits d'accès aux points de vente que les titres français en fonction de leur catégorie : IPG, CPPAP, non-CPPAP, hors presse.

Le présent amendement vise à clarifier une disposition qui, en l'état, nous semble laisser planer le doute sur l'exercice futur du droit de grève des acteurs de la distribution de la presse, comme c'est le cas au moment où nous parlons. électroniques et des postes, l'Arcep, de prononcer des sanctions contre ces acteurs lorsqu'ils feraient application de leur droit de grève dans le cadre de négociations professionnelles ? L'articulation entre cette disposition et les pouvoirs de sanction conférés à l'Arcep, dont le champ a par ailleurs été étendu par la commission, laisse planer le doute. Si tel était le cas, nous n'y serions pas favorables. Il ne s'agit bien évidemment pas pour nous de renforcer le droit de grève de ces acteurs, mais simplement de maintenir le droit existant sur cette question. Cet amendement est complémentaire de l'amendement suivant, tant ils visent tous les deux à renforcer l'équilibre entre deux principes fondamentaux à valeur équivalente dans notre droit : le droit de grève et la liberté de la presse. Quel

Il est évident que le régulateur ne pourra pas reprocher à un acteur de la distribution de la presse de ne pas assurer la continuité de la distribution si ses salariés sont en grève.

Compte tenu de leur rôle stratégique dans la diffusion, il est proposé de clarifier un peu plus l'interdiction de s'opposer à la diffusion pour les points de vente, en prévoyant qu'il est interdit d'entraver par « tous tous moyens » cette diffusion. Cette nouvelle qualification devrait permettre de sanctionner les pratiques les plus subtiles d'opposition, comme la dissimulation de numéros dont les contenus sont de nature à heurter les convictions des gérants de ces points de vente. II ne peut exister de « clause de conscience » en matière de liberté de la presse Son auteur fait évidemment référence à l'épisode, que je n'hésiterai pas à qualifier de scandaleux, du diffuseur ayant refusé de proposer un titre qui heurtait ses convictions personnelles. En ce sens, on ne peut que saluer votre démarche, ma chère collègue. Cependant, la rédaction de l'article me paraît déjà suffisamment claire sur ce point : le diffuseur ne peut pas s'opposer à la diffusion d'un titre de J'ajoute que l'épisode regrettable auquel vous faites certainement référence est un cas unique, qui a profondément choqué dans une profession justement très attachée à la neutralité. Il me paraît donc peu utile de modifier la rédaction du texte, sans changement sur le fond, d'autant qu'il sera bien difficile de qualifier ce comportement délictueux. La commission émet donc un avis défavorable.

à l'accord interprofessionnel sans en avoir pour autant à supporter les effets. Cela constitue une entrave majeure à la liberté du commerce de la presse et crée une situation de conflit d'intérêts, voire d'abus de position dominante. Compte tenu de la forte présence de la presse d'information politique générale au sein de ces organisations professionnelles, cette presse participerait ainsi à la négociation d'un accord consacré uniquement à la régulation de ses concurrents. Le présent amendement vise donc à permettre uniquement aux entreprises concernées d'être parties à l'accord, à l'inverse de la rédaction actuelle du texte, qui, je le répète, permet à tous les titres, notamment IPG, de statuer sur l'accès à des titres « commission paritaire » au réseau de distribution.

ses défauts. En étant extrêmement avantageux pour l'ensemble des publications produites en France, y compris des publications ludiques ou autres, il présentait l'avantage pour de jeunes publications de bénéficier d'un système de distribution leur permettant de toucher facilement un large prisme de lecteurs, et d'aligner les conditions de mise en concurrence des titres ainsi produits. Dans le nouveau système proposé, l'avenir des nouvelles publications pose question, notamment en matière d'IPG. Seront-elles admises à la qualification d'IPG dès le premier numéro ? L'objet de cet amendement est donc de souligner le léger recul que présente ce projet de loi du point de vue du renouvellement de la presse, en particulier de l'IPG, dès lors que les titres existant au moment de l'entrée en vigueur de la loi semblent bénéficier d'une forme de rente de position. Nous avons conscience que certains acteurs utilisent déjà la stratégie des premiers numéros pour alimenter le marché de la presse de contenus à la qualité variable. C'est pourquoi nous sommes ouverts à une rectification de notre amendement, qui permettrait de concilier l'objectif de soutien

Cette définition méconnaît un grand nombre de critères pris en compte par les nombreux titres de presse dans leur stratégie de distribution et liés à des secteurs d'activités bien particuliers. Il en est ainsi, notamment, des titres de la presse hippique et de l'information aux consommateurs. Le présent amendement vise donc à préciser

vise à exclure de la négociation de l'accord interprofessionnel qui déterminera l'assortiment des titres de presse CPPAP les entreprises de presse d'IPG. Les dispositions de cet amendement traduisent une forte méfiance de la presse simplement CPPAP envers la presse IPG. Je trouve cependant ces craintes excessives, et ce pour trois raisons. Premièrement, il est de l'intérêt de tous, y compris et peut-être surtout de la presse IPG, que les diffuseurs présentent une sélection variée et attrayante pour les clients. Pourquoi dès lors considérer que les autres titres sont des « concurrents » comme le précise l'objet de l'amendement ? Il y a plutôt complémentarité. Deuxièmement, c'est faire peu de cas des représentants des diffuseurs, qui n'ont bien entendu aucun intérêt à appauvrir leur offre et le feront savoir durant la négociation. Troisièmement, c'est également oublier le rôle central des diffuseurs eux-mêmes, qui auront toute latitude, notamment grâce à l'amendement adopté l'initiative de notre collègue Jean-Pierre Leleux, pour obtenir enfin les titres et les quantités souhaités. Il faut le dire avec force : les titres qui se vendent, comme la presse hippique ou d'association de consommateurs, seront toujours disponibles dans les linéaires. Dès lors, cet amendement, qui complexifierait fortement le système, ne me paraît pas utile.

compris dans l'accord interprofessionnel destiné à déterminer l'assortiment. Les premiers numéros ont toujours eu une place particulière. La décision du Conseil supérieur des messageries de presse, le CSMP, du 22 décembre 2011, la première sur les assortiments, et qui malheureusement n'a pas été suffisamment appliquée, prévoyait déjà un accès illimité pour les premiers Toutes les parties prenantes que nous avons pu rencontrer, en particulier Culture Presse, ont garanti que les premiers numéros auront accès au réseau et pourront trouver leur clientèle. L'amendement proposé a pour objet de garantir cet accès dans la loi. Cependant, il existe un risque, bien identifié dans la profession, qui est celui du « faux premier numéro », soit les revues essentiellement composées de publicités qui ne font que quelques numéros, disparaissent, et réapparaissent sous une autre forme presque identique. Ce risque serait majoré par cet amendement. de l'amendement n° 5 rectifié d'André Gattolin devrait permettre une présentation efficace et dématérialisée de tous les numéros aux diffuseurs. Il me paraît donc préférable de faire confiance à la négociation

Le paradoxe est que la presse hippique mentionnée ici, avec la presse de défense des consommateurs, rencontre un réel succès commercial et n'a donc bien entendu pas vocation à disparaître des linéaires. Il est donc difficile d'envisager que l'accord interprofessionnel puisse réduire sa place, bien au contraire. Cependant, le sous-amendement n° 55 du Gouvernement tend à apporter une précision utile, en prenant explicitement en compte l'actualité. Cela constitue une forme de rappel au moment de la négociation et pourra rassurer un peu certains titres. En conséquence, je suis favorable à ces deux amendements

Enfin, l'amendement n° 20 vise à constituer une commission chargée de garantir que l'ensemble des publications sera disponible dans chaque bassin de vie. Cette mesure est tout à fait louable dans son principe, mais peu applicable dans les faits. Elle suppose la définition de « bassins de vie », soit

Nous sommes très favorables à ce droit d'assortiment, qui devrait permettre de renforcer la vitalité économique des vendeurs de presse sur tout notre territoire, et ce de façon pragmatique, la faculté à chacun de choisir les titres qui lui paraissent trouver des débouchés auprès de sa clientèle. Je rappelle que, comme vous l'avez souligné dans votre rapport, mon cher collègue : « Entre 2011 et 2017, 5 300 points de vente ont été fermés, soit une baisse de 19 %. La filière estime que le réseau devrait se réduire à 21 000 points de vente en 2020, contre 23 217 fin 2017. Nous cherchons donc à anticiper les obstacles qui pourraient s'opposer à un plein exercice de ce droit d'assortiment, dans la continuité des travaux de la commission. À ce stade de nos réflexions, il nous semble que l'existence de grands groupes de presse rassemblant des titres de la presse IPG et de la presse CPPAP pourrait biaiser ces accords et conventions, dès lors qu'un grand éditeur pourrait proposer de conditionner la vente de l'un de ses titres à celle d'un ensemble d'autres titres moins attractifs.

Cet amendement tend à proscrire la pratique des ventes liées dans le cadre de l'assortiment et des conventions passées par les diffuseurs. Cette précision paraît superfétatoire. En effet, l'article L. 121-11 du code de la consommation s'applique bien évidemment à la presse-

pourra être effectuée de manière dématérialisée. La disposition prévue permet ainsi de lever une ambiguïté et de tendre vers l'objectif de simplification de l'activité des diffuseurs, qui nous rassemble tous. Quel

Cet amendement vise à éviter que deux entreprises appartenant au même groupe économique ne puissent se regrouper en une coopérative de distribution. En effet, la réduction du seuil permettant de

Cet amendement vise à introduire davantage de transparence dans les décisions concernant les possibles dérogations applicables aux barèmes et à réintroduire la faculté pour l'assemblée générale des sociétés coopératives de se prononcer sur ces possibles dérogations de la commission ? Il s'agit de rétablir la validation des barèmes par les coopératives, par un vote en assemblée générale. Le projet de loi prévoit que les barèmes sont non plus approuvés par les coopératives, mais proposés par les sociétés agréées.

Darcos. Aux termes du projet de loi, le cahier des charges devant être respecté par la société de distribution qui sollicite l'agrément sera fixé par décret au vu d'une proposition du nouveau régulateur, c'est-à-dire Afin de s'assurer que l'Arcep ait connaissance des attentes des futurs clients de ces sociétés agréées, il convient de prévoir une consultation préalable des organisations professionnelles représentatives des entreprises de presse. Quel est l'avis de

Nul ne sait quel avenir les lecteurs réservent à la presse papier devant être acheminée par véhicules vers des points de vente répartis sur l'ensemble du territoire. Sous le Second Empire, pour desservir ses 80 000 points de vente répartis sur tout le territoire, le groupe Hachette pouvait compter sur le soutien logistique des réseaux ferrés, comme l'a démontré l'historien Jean-Yves Mollier. Aujourd'hui, nous avons tous connaissance des capacités de fret ferroviaire, qui participent à l'isolement de nombreux territoires ruraux- autre cheval de bataille du RDSE. Nous nous fondons sur des estimations pessimistes quant à l'avenir du papier, dont on n'a de cesse d'annoncer la disparition prochaine. Or, dans le même temps, dans la Silicon Valley, berceau des Gafa, on observe une forme de rejet du tout numérique. Sans vouloir extrapoler, il est possible que le papier n'ait pas dit son dernier mot et que sa diffusion physique reste nécessaire pour quelques décennies encore. Dans cette optique, le présent amendement vise à inciter les sociétés chargées de la diffusion de la presse à avoir recours à des moyens de transport à faible émission de gaz à effet de serre. Tel qu'il est rédigé, il est relativement peu contraignant et relève surtout de l'incitation.

David Assouline. L'alinéa 2 du nouvel article 11 de la loi Bichet précise les modalités d'octroi de l'agrément : respect d'un cahier des charges définissant les obligations des candidats et déterminant les besoins de service fixés par décret sur proposition de l'Arcep. L'Arcep aura donc compétence pour connaître des problématiques de la distribution de la presse. Le CSA n'héritera pas d'une nouvelle compétence, pas plus que la récente Autorité de régulation de la distribution de la presse, qui aurait pu voir ses compétences et son pouvoir coercitif renforcés. Au lieu de Au lieu de cela, le Gouvernement a préféré reprendre à son compte les préconisations qui figuraient dans le rapport Schwartz, estimant que la régulation de la distribution de la presse ne nécessitait pas une instance dédiée, où, sur le plan économique, le chiffre d'affaires du secteur est inférieur à 500 millions d'euros et que, sur le plan juridique, le maintien du pluralisme est garanti par le Conseil constitutionnel. On ne voit pas sur quel fondement repose le seuil économique de 500 millions d'euros. Quant au Conseil constitutionnel, encore faut-il qu'il soit saisi pour juger des éventuelles atteintes au pluralisme qui, dans le cadre de la distribution de la presse, pourront être quotidiennes et renouvelées. Compte tenu des compétences et de la philosophie guidant l'Arcep, qui est habituée

Ces précisions paraissent très utiles, même si le Conseil d'État et l'Arcep ont mis en garde contre une définition trop précise du contenu du cahier des charges qui contraindrait en réalité la pratique de la régulation.

Afin de remplir l'objectif constitutionnel de respect du pluralisme et de libre choix des lecteurs, auquel concourt le système de distribution de la presse et que le projet de loi vise à garantir- il s'agit des nouveaux articles 4 et 5-1 de la loi Bichet, notamment -, il est essentiel que les contraintes propres à la distribution des quotidiens nationaux soient prises en compte dans le cahier des charges où sont définies les obligations des sociétés agréées pour assurer la distribution groupée des journaux. En effet, la distribution des quotidiens est soumise aux contraintes spécifiques suivantes : travail de nuit, pic d'activité, vente de l'après-midi, parution le dimanche et les jours fériés, horaires de distribution, schéma logistique propre, obligation de couverture territoriale complète.

que le cahier des charges qui subordonne l'agrément des sociétés habilitées à opérer la distribution groupée prévoit une distribution des quotidiens sur la totalité du territoire. Quel est l'avis de la commission ? Cet amendement vise à préciser que l'agrément tient compte des contraintes techniques liées à la distribution des quotidiens.

Il est urgent d'établir une continuité des obligations s'imposant aux organismes de presse, que celle-ci soit diffusée par papier ou par voie numérique. L'interprétation actuelle des normes européennes conduit à un système à deux vitesses.

les services en ligne, notamment les réseaux sociaux, aucune de ces règles n'est garantie. Ces derniers ne sont pas soumis à l'obligation d'assurer le pluralisme et d'offrir des conditions plus favorables de distribution aux titres de presse IPG.

tendant à mettre en avant des contenus similaires à ceux que plébiscitent les utilisateurs, quelle que soit leur qualité. Par cet amendement, nous voulons signifier au Gouvernement qu'il est urgent d'agir, alors que plane la menace de manipulation d'utilisateurs par des puissances étrangères, dans un contexte électoral. En outre, l'étude d'impact fait état d'une jurisprudence européenne favorable, des droits de l'homme, et des précautions prises parfois par le législateur européen en faveur du pluralisme et de la protection de la liberté de la presse. La directive e-commerce régulièrement invoquée date de 2004. À cette époque, les réseaux sociaux qui influencent aujourd'hui nos concitoyens n'existaient pas ou n'avaient pas développé une telle pratique de mise en avant de contenus de presse. C'est pourquoi nous pensons que des dispositions nationales sans attendre un mouvement européen, lequel pourrait être long compte tenu des divergences de vues entre États membres sur la question du pluralisme ... Nous sommes confiants sur l'issue d'un bras de fer devant les juridictions européennes et nous estimons qu'il est plus qu'urgent d'agir en faveur de notre démocratie. Quel

mais aussi dans le partage de la valeur entre les différents acteurs du secteur considéré, en l'occurrence la presse. C'est tout l'enjeu des droits voisins ou droits d'auteur, par exemple, pour les éditeurs de presse. La parole est à Mme la présidente de la commission.

Mais il est bon que nous fassions vivre ce débat. Il est très important que nous obtenions la réouverture de la directive e-commerce, et ce pour maintes raisons.

a plus de quinze ans, ce qui représente un centenaire à l'échelle du développement des nouvelles technologies ! Comment continuer à s'y conformer sans l'adapter à la nouvelle réalité de son champ d'application ? Les dispositions du projet de loi sur les kiosques numériques nous paraissent aller dans le bon sens. En matière de plateformes numériques, si le texte comporte certaines avancées en termes de transparence, nous les jugeons néanmoins insuffisantes.

préciser que, en dépit de ces préférences, les informations fournies respectent le pluralisme. Un tel schéma est en réalité technologiquement complexe. Il impose une forme de modèle à des opérateurs privés et il pose de nouveau la question des limites autorisées par le droit communautaire, voire le droit commercial. La commission émet

je suis l'auteur. Cela étant, afin d'assurer l'efficience de l'extension des principes de la loi Bichet à la diffusion numérique et de garantir ainsi la réelle sauvegarde du pluralisme de la presse d'information politique et générale en ligne, il convient de compléter les dispositions du projet de loi sur la diffusion numérique sur plusieurs points. opérer un renforcement des conditions de mise à disposition des titres IPG par les services en ligne. Certains acteurs de la distribution numérique groupée proposent des modèles de rémunération peu avantageux, voire sans réel partage de la valeur- Apple News conserverait plus de 50 % des revenus issus de la presse -et peu transparents pour les éditeurs- la traçabilité de la diffusion n'est pas toujours certifiée par un tiers. Pour être efficace, l'extension des principes de la loi Bichet à la diffusion numérique doit permettre de rééquilibrer les rapports commerciaux entre les plateformes et les éditeurs de la presse IPG en veillant, d'une part, à l'image du dispositif sur le prix unique du livre numérique, à ce que les conditions techniques et financières de reprise des titres IPG par les plateformes soient raisonnables pour l'éditeur de presse, d'autre part, à ce que les conditions de reprise soient acceptables de sorte que l'autorité de régulation compétente puisse veiller, comme pour la diffusion imprimée, à une juste répartition de la chaîne de valeur entre les parties prenantes. Il convient ensuite de valoriser les contenus en créant une labellisation « Presse d'information politique et générale Pour assurer l'objectif de défense du pluralisme de la presse IPG et surtout pour garantir le libre choix des lecteurs dans la profusion des contenus disponibles en ligne, il est nécessaire de prévoir des mesures de visibilité et de promotion de l'accès à la presse IPG. Tel est l'objet de l'amendement n° 7 rectifié, qui répond en grande partie aux

le présent amendement vise à atténuer la distinction entre diffusion numérique et diffusion papier. Le projet de loi confie le contrôle du respect des obligations de diffusion numérique à la DGCCRF,

n° 7 rectifié vise à promouvoir la mise en avant, sur les kiosques numériques et les plateformes, des contenus issus de la presse en ligne d'information politique et générale, grâce à un label « Presse d'information politique et générale ».

comme nous l'avons dit lors du débat sur la proposition de loi relative à la lutte contre la manipulation de l'information. Le fait de singulariser la presse IPG pourrait de plus être mal perçu par les autres presses, qui s'estimeraient discriminées. Par ailleurs, il serait préférable que cette initiative émane des acteurs eux-mêmes, plateformes et éditeurs, afin de de parvenir à une application consensuelle et efficace. Dès lors, tout en reconnaissant la légitimité de cette interrogation, j'émets un avis défavorable sur cet amendement. 48 rectifié vise à unifier la régulation de la presse sous l'égide de l'Arcep. La question posée est tout à fait légitime, mais il n'existe pas de solution simple, chère Françoise Laborde. D'un côté, la DGCCRF est compétente pour la régulation des plateformes en ligne,

j'incline à penser qu'il vaut mieux avoir, à ce stade, un régulateur unique pour les plateformes, qui serait donc la DGCCRF. De plus, le projet de loi confie déjà beaucoup de compétences à l'Arcep. Il ne me paraît pas opportun d'aller plus loin. En conséquence, j'émets un avis défavorable sur cet amendement.

financière du système, mais également la méfiance généralisée qui mine les relations entre les éditeurs. Dès lors, la proposition d'instaurer un régulateur indépendant me paraît très raisonnable. Elle fait d'ailleurs consensus dans la profession. Je propose donc de donner sa chance à l'Arcep, et j'émets un avis défavorable sur cet amendement.

aient attiré l'attention à de multiples reprises sur le fait que cette concurrence était mortifère pour le secteur. Les différents gouvernements n'ont jamais agi alors qu'il

Les articles 15 et 16 de la loi de 1947, modifiés par l'article 1, définissent le nouveau champ de compétences de l'Arcep en matière de distribution de la presse, en lui confiant une compétence générale de régulateur du secteur. du secteur. Aux termes de la loi, les compétences de l'Arcep ne s'étendent pas à la régulation du marché de la distribution des éditeurs de presse locale qui, depuis 1947, s'inscrit hors de la logique de groupage.

Laborde. Le présent sous-amendement vise à intégrer le respect du pluralisme à la nouvelle mission de régulation du secteur de la distribution de la presse incombant à l'Arcep. Certains observateurs considèrent en effet que, compte tenu de ses champs d'intervention traditionnels, l'Arcep ne serait pas le meilleur acteur pour mener à bien cette mission de gouvernance. tend à lever ces inquiétudes en orientant la mission de l'Arcep, non seulement vers des objectifs économiques, mais également vers l'objectif qualitatif de préservation du pluralisme. Comme nous l'évoquions lors de la discussion générale, la distribution de la presse n'est pas un secteur économique comme les autres,

On peut penser que la régulation de la presse, au sens de la loi de 1947, modifiée par le présent projet de loi, vise bien la presse recourant à la distribution groupée, en application notamment de l'article 3

à M. David Assouline. Aux termes du projet de loi qui nous est soumis, les barèmes ne seront plus votés par l'assemblée générale des coopératives comme précédemment. Les sociétés agréées devront les soumettre à l'Arcep sans aucune obligation de communication publique. On ne connaît que trop les dérives d'une telle absence de transparence, qui a précédemment permis aux éditeurs de négocier, malgré les barèmes ainsi votés, des conditions privilégiées avec une société de messagerie qui n'avait pas les moyens juridiques d'opposer un veto à de telles demandes.

dispositions du projet de loi prévoyant que les sociétés de distribution agréées n'auront plus de liens capitalistiques avec les coopératives devraient permettre de mettre fin au système pervers de ristournes sur les barèmes consenties aux éditeurs, à la fois clients et actionnaires sociétaires des messageries. Ce système pervers faisait que l'intérêt du client à obtenir une ristourne contrevenait à ce qu'aurait dû être celui du sociétaire, et surtout celui de la société de messagerie. Il ne devrait donc plus y avoir d'obstacle majeur à maintenir des barèmes cohérents et correspondants aux prestations réelles. Néanmoins, je tiens à ce que la législation incite à la cohérence des barèmes et, pour satisfaire cet objectif, rien ne vaut la transparence, qui passe par la publication de ces de ces barèmes. Cet amendement tend donc à donner compétence à l'Arcep pour rendre publics les barèmes, au même titre qu'elle rendra public le schéma territorial, qui mentionnera les distributeurs centraux de presse. L'Arcep n'aura aucune difficulté à honorer cette nouvelle mission, puisqu'elle aura, en vertu de la loi modifiée, été informée par les sociétés agréées de leurs conditions tarifaires et qu'elle aura même pu les inciter à les réviser, voire à les encadrer de façon pluriannuelle. Quel est l'avis de

les éléments les plus importants de ces derniers le seront également. À tout le moins, le respect des grands principes de la loi serait vérifié. Cet avis de l'Arcep pourrait toutefois être utilement complété par la publication des barèmes qui permettrait en particulier d'apporter un degré de transparence inédit à la distribution de la presse. En conséquence,

Quel est l'avis de la commission ? Cet amendement vise à revenir au texte initial du projet de loi en rétablissant le caractère d'orientation du schéma territorial de distribution mentionnant les dépositaires centraux. la commission a adopté un amendement pour supprimer ce caractère d'orientation. Comme je l'avais alors expliqué, il s'agit, sans revenir sur l'avis du Conseil d'État ou de l'Arcep, de ne pas négliger ces acteurs importants et vertueux du système que sont les dépositaires centraux.

Monsieur le ministre, vous avez mis en avant la réelle plus-value qu'apporte la profession des dépositaires de presse par rapport à une simple distribution de titres de presse. En effet, ces entreprises n'ont pas qu'une fonction strictement logistique ; elles ont aussi une mission financière et commerciale d'accompagnement des diffuseurs et d'animation du réseau au quotidien. Le projet de loi que nous examinons aujourd'hui ne rend pas suffisamment compte de l'importance du rôle des dépositaires, et il est totalement silencieux sur leurs conditions d'exploitation et d'encadrement de leur activité.

; ils n'ont aucunement démérité dans les missions qui leur ont été confiées, et ils ont investi des fonds personnels pour permettre la restructuration de la distribution régionale, sans jamais bénéficier d'aides de l'État. Sans aucune aide, ces professionnels ont réussi, par la mutualisation des flux de l'ensemble des produits de presse, à assurer de façon constante et efficace la distribution pour la partie la plus sensible des opérations, à savoir le dernier kilomètre. C'est ce système qui permet aujourd'hui aux marchands de journaux d'avoir un interlocuteur unique et de proximité pour la gestion de leur activité presse. En outre, en traitant de manière exhaustive les magazines et quotidiens nationaux, les dépositaires sont un des piliers de la neutralité de la distribution, objectif que le législateur vise depuis 1947. Ils font ainsi vivre le pluralisme et la diversité de la presse sur l'ensemble du territoire, y compris dans nos campagnes et nos villages les plus difficiles d'accès.

commission ? Cet amendement, avec celui du Gouvernement, soulève la question des dépositaires centraux, qui constituent le niveau 2 de la distribution. Il convient de rappeler que ce niveau 2 n'est pas rendu obligatoire par la loi Bichet en vigueur, qui précise juste, en son article 18-6, le CSMP, fixe leurs règles d'organisation et missions. La pratique en a cependant fait un élément incontournable, de surcroît apprécié de tous. Les dépositaires centraux sont majoritairement des indépendants, qui ne se limitent pas à la fonction logistique et financière, mais qui jouent également un rôle d'animation de réseaux. Toutefois, et alors que le projet de loi qui nous est proposé place au centre de la distribution des sociétés agréées, qui devront être les plus efficaces possible, il ne paraît pas opportun de figer dans le marbre de la loi l'organisation actuelle. Le Conseil d'État a d'ailleurs été très clair sur ce point. Je suis cependant persuadé que les sociétés agréées auront tout intérêt à se rapprocher des dépositaires centraux. L'avis de la

avec ces accords interprofessionnels et ces accords de gré à gré pour les titres non CPPAP entre les marchands de journaux et les éditeurs de presse.

de la performance et de la compétence des dépositaires de niveau 2, je suis certain qu'ils saisiront toutes les opportunités pour améliorer encore la qualité de ce réseau de dépositaires de presse.

est ainsi désignée comme garante de la liberté de distribution de la presse. Toutefois, en retenant une terminologie générale de distribution de la presse pour définir le champ de compétence de l'Arcep, le texte des articles 15 et 16 semble étendre le contrôle de l'Arcep à l'ensemble de la distribution imprimée, en incluant l'auto-distribution organisée par une entreprise de presse. Or ce mode de distribution s'inscrit,

ne vise pas à remettre en question le système d'auto-distribution pratiqué avec efficacité par la presse quotidienne régionale ni à confier à l'Arcep sa régulation. Il convient donc, pour préciser cette intention du Gouvernement, d'écrire dans la loi que les compétences de l'Arcep ne s'étendent pas à la régulation du marché de la distribution des éditeurs de presse locale. Ces précisions s'inscrivent dans la

Au demeurant, les régulateurs n'ont jamais revendiqué de compétences concernant la presse locale auto-distribuée. Afin de lever toute ambiguïté, il convient ainsi de préciser dans la loi que le champ de compétence de l'Arcep, s'agissant de la régulation de la presse imprimée, se limite à la distribution groupée de journaux et de publications. Par voie de conséquence, les dispositions qui confient de nouveaux pouvoirs, notamment de sanction, à l'Arcep sont mises en cohérence avec la réduction du champ d'intervention de celle-ci à la distribution groupée. Mes chers collègues,

Il faut donc veiller à un juste équilibre entre défense du pluralisme et respect des droits des diffuseurs de presse. C'est pourquoi il est important de le préciser et de s'assurer des droits et responsabilités de tous les acteurs.

semble toutefois manquer de clarté. Les pouvoirs de sanction de l'Arcep sont déjà prévus pour les entreprises de presse, les sociétés coopératives et les sociétés agréées, ainsi que les kiosques numériques. On ne voit pas bien qui sont les autres personnes ou entreprises impliquées dans la distribution. Pour cette raison, j'émets un avis défavorable

en cas de manquement aux obligations légales, l'Arcep peut sanctionner l'auteur de ce manquement après une mise en demeure prononcée dans un certain délai. Le texte précise que ce délai est d'un mois ou moins, ou moins, selon la gravité du manquement. Toutefois, au regard de la particulière gravité de l'opposition à la diffusion d'un titre de presse, il est proposé de un délai dérogatoire plus adapté à ce manquement particulier. Le présent amendement vise un délai réduit de vingt-quatre heures, compte tenu de la durée de vie économique particulièrement courte d'un quotidien. Constater, plus d'un mois après sa parution, l'obstruction à sa diffusion n'aurait pas grand sens. Quel ? Cet amendement vise à fixer un délai plus bref en cas de manquement aux obligations de distribution d'un titre de presse d'information politique et générale. Il tend donc à instaurer une protection spéciale pour les cas où la distribution d'un titre de presse IPG serait menacée.

Comme l'amendement précédent, et dans l'esprit du travail opéré par le rapporteur, cet amendement vise à étendre la palette d'instruments à disposition de l'Arcep, afin de lui permettre de prononcer des astreintes dès la mise en demeure. Cela a été dit à de nombreuses reprises : la presse écrite se porte mal, et tous les manquements à des obligations conventionnelles ou légales de nature à fragiliser davantage des titres de presse devraient être sanctionnés le plus fermement possible. Les juristes sont unanimes sur l'efficacité de l'astreinte comme instrument pour la mise en oeuvre d'une décision. Compte tenu de la procédure relativement longue de sanction prévue par le texte, avec une première mise en demeure, puis une sanction en cas de non-respect de la mise en demeure, doter l'Arcep d'une prérogative d'astreinte pourrait lui être très utile. Quel est l'avis de

car elle va dans le sens du texte et crédibilise le dispositif de régulation. Introduire une astreinte journalière au stade de la mise en demeure de la procédure, c'est-à-dire avant que la formation restreinte de l'Arcep se soit saisie du sujet,

Il s'agit de doter les maires, y compris ceux des territoires ultramarins, d'un outil concret de préservation de la vitalité des centres-villes, en leur permettant de s'opposer effectivement, et bien entendu au cas par cas, à l'implantation des points de presse dans les zones commerciales hors de la ville, lorsque cette implantation est de nature à dévitaliser le centre de la commune.

par le texte. Nous pensons qu'il faut traiter la question de leur statut, notamment reconnaître qu'ils sont réputés salariés à partir du moment où ils exercent leur activité dans des conditions de droit ou de fait caractérisant un lien de subordination juridique vis-à-vis d'une autre personne physique ou morale. Quel est l'avis de

Il convient de préciser que la fin de l'insécurité juridique dans laquelle ils sont plongés a été négociée avec eux et les éditeurs, afin de développer le portage de presse. L'avis de la commission est Une fois de plus, M. le rapporteur a été très clair. L'article 6 sécurise juridiquement la situation des VCP. Je rappelle qu'ils exercent souvent leur activité de portage en complément d'une autre activité. C'est alors pour eux un revenu d'appoint, et non une activité à temps plein. Je crois vraiment qu'il ne serait pas judicieux de remettre en cause leur statut de travailleur indépendant, car cela risquerait de décourager le recours au portage, qui est pourtant un élément incitatif pour que le lectorat s'abonne à des publications. Je suis défavorable

pour le portage de toute la presse, sous réserve que le portage, hors presse IPG, soit effectué à titre accessoire, les porteurs salariés ne continueront à bénéficier de ces exonérations que pour les quotidiens et les hebdomadaires IPG au sens de l'article 39 du code général des impôts. Il en résulterait donc un périmètre d'exonérations sociales plus large pour le portage VCP par rapport au portage salarié, ce dernier restant limité aux seuls quotidiens et publications hebdomadaires IPG à diffusion locale. Or à l'heure où l'offre de portage sur tout le territoire doit permettre de consolider la filière de la distribution de la presse et être accessible à tous les éditeurs, quels que soient leur famille de presse ou le modèle de portage choisi, il me semble qu'un traitement égalitaire doit être assuré entre tous les réseaux de portage. Le Gouvernement poursuivant une logique d'harmonisation des dispositifs relatifs au portage, il devrait donc lui importer que tous les exemplaires papier puissent être distribués selon les mêmes conditions par tous les réseaux de portage, qu'ils emploient des salariés ou qu'ils mandatent directement ou indirectement des VCP. Dès lors, et pour éviter toute problématique logistique ou tout déséquilibre économique entre les acteurs, l'amendement vise à aligner les bases de cotisations pour tous ceux, salariés ou VCP, qui distribuent la presse par portage.

Sur ce sujet très technique et très complexe, je souhaiterais des éclaircissements : monsieur le ministre, vous paraît-il nécessaire d'aligner les deux régimes et quel en serait le coût ?

au jour. Comme je veux vraiment soutenir le combat que va devoir maintenant mener M. le ministre de la culture auprès de beaucoup

De toute façon, les parlementaires socialistes qui siègent à l'Assemblée nationale prendront le relais si la promesse n'est pas tenue, pour redire que le principe d'égalité de traitement

Beaucoup de points ont été modifiés, précisés, et ce texte est de plus en plus acceptable.

j'ai le sentiment que beaucoup espèrent achever le malade Presstalis. Et si tel est le cas, c'est tout de suite que l'on ira chercher quelqu'un d'autre, car il n'y aura alors plus personne pour distribuer la presse dans le pays.

date. Il paraît certain que le cahier des charges et les premiers agréments ne seront délivrés que quand les acteurs historiques auront pu se mettre au niveau, ce qui, j'en suis

car il n'y aura plus personne pour distribuer la presse. Je ne veux pas de ce scénario. C'est peut-être un scénario catastrophe, mais, vous le savez, mes

Presstalis est en très grande difficulté. Les grandes plateformes et les grands acteurs numériques de la logistique sont-ils prêts à jouer le jeu

pour s'adosser à des entreprises spécialistes de la logistique, soit pour nouer des partenariats très particuliers avec ces entreprises. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons ce texte. ce texte. M. le rapporteur a raison : il faut donner la possibilité malgré tout à l'État de réagir en cas de bouleversement considérable dans la distribution de la presse. Cependant, je le redis une troisième fois devant vous, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, l'objectif du Gouvernement est d'ouvrir

vote. Le groupe socialiste et républicain se réjouit d'avoir pu amender le projet de loi relatif à la modernisation de la distribution de la presse, qui sortira ainsi du Sénat avec des améliorations substantielles. Nous les devons au rapporteur et à d'autres collègues présents dans l'hémicycle.

Il est satisfaisant que les principes de la loi Bichet de 1947 soient maintenus : système coopératif, liberté de distribution, égalité de traitement guideront toujours la distribution des journaux. Il était urgent d'agir pour tenter d'enrayer la fermeture des points de vente de presse, ce que ce en partie liée, il est vrai, à la chute des ventes de la presse papier au profit de la presse numérique. Il était également nécessaire de mettre un terme au système hérité de 1947, qui faisait des éditeurs de presse à la fois des actionnaires et des clients des messageries, entraînant des conflits d'intérêts qui se concrétisaient par des ristournes systématiques accordées aux plus gros. Ces ristournes ont causé la perte financière des messageries, et plus particulièrement de Presstalis. Il faut espérer que le nouveau système d'agrémentation des sociétés de distribution, qui distribueront la presse de façon groupée, par l'Arcep, tiré d'une nouvelle compétence de régulateur de la distribution, permettra de clarifier le secteur. Néanmoins, le choix de cette autorité, qui ne raisonne normalement qu'en termes économiques et non au regard de l'objectif constitutionnel du maintien du pluralisme, laisse les sénateurs socialistes perplexes. Par ailleurs, nous nous réjouissons d'avoir pu améliorer le dispositif en votant les amendements du rapporteur et en Ils concernaient l'encadrement des pouvoirs dont disposera l'Arcep en termes de garanties du maintien du pluralisme, de meilleur maillage du territoire, de transparence des tarifs pratiqués. Nous sommes aussi contents d'avoir limiter le champ d'intervention de l'Arcep à la seule distribution groupée de la presse, afin que les éditeurs qui s'auto-distribuent, principalement la PQR, puissent continuer à le faire, sans droit de regard de cette autorité. Il faut conclure ! Face à l'équilibre fragile auquel aboutit le projet de loi, les sénateurs du groupe socialiste et républicain ont

et la réalité. Nous prenons acte des engagements sur les principes et nous ne prenons pas à la légère les paroles prononcées en la matière.

la rupture du service de la distribution de la presse résonnerait comme une catastrophe démocratique majeure. La question est donc extrêmement sérieuse.

améliorer l'existant. Le système de distribution de la presse avait besoin d'être modernisé et il le sera grâce au texte de la commission. Le rapporteur a présenté